Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Yves Roux, auteur de la proposition de loi. Monsieur Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui s'inscrit au coeur des missions institutionnelles du Sénat. Le sujet du désenclavement n'est en rien nouveau, mais il revêt aujourd'hui une acuité toute particulière. Les grands débats qui se déroulent en ce moment dans toute la France l'ont remis à l'ordre du jour de manière plus aiguë encore, parfois plus douloureuse,

Plus que jamais, nous avons besoin d'un cadre et d'un socle national qui garantissent le développement équilibré de nos territoires, maintenant et pour le futur. C'est la raison pour laquelle nous avons saisi cette occasion, avant même la discussion du projet de loi d'orientation des mobilités, d'inscrire dans la loi un objectif national de désenclavement.

en compte la réalité d'une France polycentrée, dont les territoires ont vocation à assurer, dans la perspective d'un enjeu environnemental majeur, leur propre trajectoire de développement durable.

aucune partie du territoire français métropolitain continental ne [serait] située à plus de 50 kilomètres ou de 45 minutes d'automobile soit d'une autoroute ou d'une route expresse à 2x2 voies en continuité sur le réseau national, soit d'une gare desservie par le réseau ferré à grande vitesse

Madame la ministre, nous connaissons les lieux à désenclaver, pour lesquels la solidarité nationale doit s'exercer. Nous connaissons aussi votre souhait de privilégier les transports du quotidien. Les citoyens et les élus qui les représentent ont désormais besoin de garanties claires inscrites dans la loi. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. J'en viens au texte même. Notre proposition de loi vise à améliorer l'accès aux infrastructures routières, ferroviaires et aériennes dans les territoires identifiés comme prioritaires. La route constitue à cet égard le moyen universel de déplacement dans ces territoires. J'ai grand plaisir à prendre les transports en commun en venant à Paris, mais force est de constater que certains modèles ne sont pas exportables.

depuis presque trente ans, les élus des Alpes-de-Haute-Provence bataillent pour que leur ville préfecture- excusez du peu ! -soit reliée à l'autoroute ...

Nous proposerons, par voie d'amendement, sur l'initiative notamment de mon collègue Jean-Pierre Corbisez, de préciser ces distances en intégrant la notion de distance parcourue par rapport à la ville préfecture, lieu de référence commun à toute la ruralité. L'article 2 prévoit d'inscrire dans la loi un principe d'adaptation s'imposant à l'État, en vue de prendre en compte des projets plus adaptés aux réalités topographiques, économiques et financières.

Je rappelle ici que le désenclavement aérien est censé être assuré par une couverture aérienne minimale. Les entreprises de transport concernées sont soumises à des obligations de service public et perçoivent des subventions à ce titre. concrètement, ces entreprises affectent du matériel ancien à ces lignes et ne parviennent pas à respecter leurs obligations. Il convenait donc à la fois de mieux contrôler le respect de ces obligations et de mieux sécuriser les financements.

L'article 5, remanié par la commission, prévoit, à l'instar de l'article 2, d'adapter l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 kilomètres par heure, avec pragmatisme et responsabilité. Nous avons déjà eu quelques débats sur dans notre hémicycle. Force est de constater que le dossier n'est pas clos et que des aménagements sont possibles. La commission a ainsi proposé que le préfet et le président du conseil départemental puissent déroger à cet objectif national uniforme de 80 kilomètres par heure, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

Elle se fonde sur une conception rénovée et moderne de l'aménagement de la France métropolitaine. Avec la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires,

Nous sommes convaincus que les enjeux liés au réchauffement climatique plaident en faveur de déplacements plus courts, plus sobres, et que nos propositions donneront corps à cette exigence.

Comment ne pas rappeler que la colère qui s'exprime aujourd'hui s'est cristallisée, au départ, sur l'augmentation de la fiscalité sur les carburants, pénalisant ceux qui utilisent en premier lieu leur véhicule pour se déplacer, c'est-à-dire, majoritairement, ceux qui n'ont pas accès à une offre de transports publics pour leurs trajets du quotidien. Le manque de solutions de transport, c'est ce que vivent tous les jours ceux qui habitent dans des territoires enclavés. Il résulte d'une offre de mobilité insuffisante, notamment en matière de transports collectifs, mais aussi d'un manque d'infrastructures de transport adaptées, soit parce que ces infrastructures sont trop lointaines, soit parce qu'elles ne sont pas aménagées pour permettre une circulation rapide. Pour répondre à cette difficulté, la proposition de loi prévoit trois axes d'action principaux. Le premier volet porte sur les infrastructures de transport. La proposition de loi vise à faire du désenclavement des territoires l'un des piliers de la programmation de ces infrastructures, c'est-à-dire un véritable critère d'analyse. elle prévoit que, d'ici à la fin de l'année 2025, aucune partie du territoire français métropolitain ne devra être située à une distance trop importante d'un centre urbain ou économique ou d'une voie de circulation rapide. En commission, nous avons ajouté un critère de distance à une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Il est en effet indispensable que l'objectif de désenclavement du territoire soit intégré dans la politique d'aménagement du territoire, c'est-à-dire dans les documents de planification de l'État et des collectivités, en particulier dans les contrats de plan État-région, comme étant un objectif prioritaire, comme l'a souligné en commission notre collègue Michel Vaspart. Il n'est nul besoin de rappeler que, par le passé, les choix en matière d'investissements ont porté prioritairement sur la réalisation de grandes infrastructures de transport, certes nécessaires, mais onéreuses, au détriment de l'entretien et de l'aménagement des réseaux existants, qu'il s'agisse du réseau routier ou du réseau ferroviaire. Vous nous direz sûrement, madame la ministre, que le gouvernement auquel vous appartenez a décidé d'infléchir cette tendance- vous l'avez d'ailleurs rappelé hier lors des questions d'actualité au Gouvernement, en répondant à M. Éric Gold -et que le projet de loi d'orientation des mobilités que nous examinerons le mois prochain au Sénat apportera des réponses à la problématique du sous-investissement dans les infrastructures de transports du quotidien. Certes, nous ne pouvons pas nier qu'un changement d'approche, en matière de financement des infrastructures, est intervenu. Pour autant, il nous paraît nécessaire d'inscrire des objectifs de désenclavement dans le marbre de la loi, d'en faire un critère de sélection, sinon ils passeront toujours au second plan dans les politiques d'investissements et risqueront même de servir de variable d'ajustement, dans un contexte où plane une grande incertitude sur le financement pérenne des infrastructures. La proposition de loi prévoit, par ailleurs, que l'État devra veiller à adapter les infrastructures et leurs aménagements aux territoires et à leurs caractéristiques. Il s'agit, en cela, de faciliter la construction d'infrastructures routières moins lourdes, et donc moins coûteuses, dans les zones enclavées. Il n'est bien évidemment pas question de construire des autoroutes ou des routes à 2x2 voies sur tout le territoire. Le désenclavement peut passer par l'aménagement d'une route existante afin de permettre une circulation plus rapide et de répondre à la demande des habitants du territoire concerné. Le deuxième volet de la proposition de loi concerne le désenclavement des territoires par la voie aérienne. Aujourd'hui, dans de nombreux territoires, en l'absence de TGV ou d'autoroute, seule une liaison aérienne permet une connexion rapide avec les grands centres urbains, Paris et les grandes métropoles. Lorsque l'équilibre économique d'une desserte n'est pas assuré, la puissance publique peut organiser des liaisons aériennes soumises à des obligations de service public et verser, avec les collectivités et les chambres consulaires, des subventions d'équilibre aux compagnies exploitant ces lignes. De telles liaisons sont essentielles au désenclavement des territoires et sont souvent indispensables au maintien et au développement des activités économiques. Or, depuis la loi Or, depuis la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, qui a revu la répartition des compétences entre les collectivités territoriales, seuls l'État et les régions sont compétents pour organiser ces liaisons. Les autres collectivités territoriales, notamment les départements, ne peuvent le faire que par délégation des régions, s'agissant des liaisons intrarégionales, ou de l'État, s'agissant des liaisons interrégionales.

Quant aux régions, elles ne sont pas le seul échelon pertinent pour appréhender la problématique du désenclavement et y répondre. C'est pourquoi j'aurais souhaité déposer un amendement visant à donner aux départements et aux EPCI la compétence pour organiser eux-mêmes des liaisons d'aménagement du territoire,

La proposition de loi vise d'ailleurs à renforcer ce contrôle, en prévoyant que les compagnies aériennes devront transmettre aux autorités publiques des informations sur le fonctionnement des lignes de manière plus fréquente et plus transparente. Enfin, le troisième et dernier volet de la proposition de loi concerne la limitation Certes, madame la ministre, cette question ne relève pas, en tant que telle, de la problématique du désenclavement des territoires. Cependant, il est légitime qu'elle soit abordée dans ce texte, car elle a contribué au sentiment d'abandon des citoyens vivant dans les territoires ruraux que j'évoquais en introduction.

Pourtant, le Gouvernement aurait pu procéder différemment. Avant l'entrée en vigueur de la mesure, de nombreux départements ont demandé que cette décision soit décentralisée, afin qu'elle puisse être adaptée aux spécificités de chaque territoire.

Lors de l'ouverture du grand débat national, le 15 janvier, le Président de la République lui-même a indiqué être ouvert à des aménagements. Tel est le sens de l'amendement que nous avons adopté en commission à l'article 5. Il vise à donner aux présidents de département et aux préfets

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la question du désenclavement, soulevée par cette proposition de loi, est au coeur de mes préoccupations depuis plus d'un an et demi. Effectivement- les Assises nationales de la mobilité ont permis d'en faire le constat -, trop de territoires et de citoyens se sentent laissés à l'écart, oubliés des politiques publiques.

le réseau routier se dégrade et les projets de désenclavement se font attendre. En outre, une large partie de notre territoire est abandonnée au « tout-voiture moi aussi qu'il est nécessaire de répondre au sentiment d'abandon d'une partie de nos territoires et de nos concitoyens. Je porte en outre la volonté de proposer des solutions de mobilité à tous. C'est bien le coeur du projet de loi d'orientation des mobilités que nous discuterons très prochainement. En complément de l'approche de la proposition de loi, centrée sur les infrastructures, il me semble nécessaire de prendre en compte les services offerts. De même, au-delà des objectifs de développement des infrastructures, il ne faut pas perdre de vue l'enjeu lié à l'état des réseaux.

C'est la raison pour laquelle la priorité des priorités, dans la programmation des infrastructures que nous discuterons très bientôt, c'est l'entretien et la régénération. Les crédits dédiés augmenteront de 31 % sur la décennie 2018-2027 et de 25 % pour ce seul quinquennat.

Dans de nombreux territoires, l'accessibilité d'une ville, son attractivité pour les entreprises, les services de santé, les commerces va dépendre de la qualité et de la performance d'une route. Partout à travers le pays, de nombreux territoires attendent une amélioration de la qualité des routes, nécessaire à leur désenclavement, et constatent la lenteur des travaux. Même si ces routes supportent des trafics modérés, le Gouvernement considère qu'elles sont essentielles pour l'aménagement du territoire. Il est devenu nécessaire et urgent d'agir. L'État prévoit donc de promouvoir des opérations sur une vingtaine d'itinéraires de désenclavement routier au sein des contrats de plan État-région, pour un montant de 1 milliard d'euros sur dix ans. Ces opérations permettront d'améliorer les déplacements du quotidien, et donc la qualité de vie des habitants des territoires concernés. Ce sont des aménagements concrets tels que des déviations courtes, des contournements d'agglomération, des créneaux de dépassement, des rectifications de virages ou des aménagements de carrefours. Il s'agit non pas de couvrir notre territoire de routes à 2x2 voies, mais de réaliser des aménagements adaptés aux besoins, permettant de fiabiliser les temps de parcours, d'améliorer la sécurité routière et le cadre de vie des habitants. Cette démarche s'inscrit dans une politique globale de cohésion des territoires reposant sur l'ensemble des modes de transport : modernisation du réseau ferroviaire, sur les lignes structurantes comme de desserte fine, liaisons aériennes d'aménagement du territoire

Concernant l'article 3, la loi confère déjà implicitement aux départements et aux communes, ainsi qu'à toute personne publique intéressée, le droit de participer au financement des liaisons aériennes d'aménagement du territoire et des exploitants d'aéroports, sous réserve du respect de certaines règles. Une note méthodologique est d'ailleurs en cours de préparation entre le ministère de la cohésion des territoires et le ministère des transports afin de clarifier le droit existant sur ces questions de compétences et de financement.

Je suis bien consciente que, aujourd'hui, la qualité de service n'est pas satisfaisante. Je suis tout aussi agacée que vous par le niveau de qualité de service sur ces liaisons ces dernières années. Cette situation est d'autant plus contrariante que de l'argent public est mobilisé. De fait, depuis 2017, HOP !, pour l'appeler par son nom, est confrontée à des difficultés d'exploitation récurrentes sur l'ensemble de son réseau. Il est bien sûr primordial de redresser la qualité de service ; je suis fortement mobilisée sur ce J'avais demandé en juin 2018 un plan d'action à HOP !, qui a permis des améliorations notables. Le nombre d'annulations sur le périmètre des liaisons radiales exploitées par HOP

Vous le savez, HOP ! vient d'être réintégrée sous le nom Air France-KLM, ce qui réaffirme son appartenance au groupe. Je sais que le nouveau directeur général d'Air France-KLM est pleinement conscient de la nécessité d'améliorer la qualité de service sur les liaisons ailleurs, je vous rappelle que les modalités de suivi de l'exploitation subventionnée s'inscrivent dans le cadre contractuel conclu avec la collectivité ou la personne publique intéressée. Elles reposent sur une vérification du respect des obligations de service public et des équilibres économiques de la ligne. Des pénalités financières ou des amendes administratives peuvent être appliquées pour tout manquement aux obligations de service public. Au demeurant, ces liaisons sont remises en concurrence régulièrement. On peut espérer qu'un nouvel opérateur ou que le même opérateur, sous sa nouvelle direction, pourra améliorer la situation.

Cela dit, je me dois de rappeler que la mise en oeuvre de cette mesure est à placer en regard du bilan de la mortalité routière, qui ne baissait plus. L'objectif de sécurité routière ne doit pas être oublié. L'évaluation était prévue, dès le départ, au début de l'année 2020. C'est l'un des sujets discutés dans le cadre du grand débat, dont il ne faut pas préempter les conclusions. J'ajoute que, si le dispositif devait être adapté, il conviendrait naturellement de ne pas relâcher nos exigences en matière de sécurité routière. L'une des difficultés de nos territoires, qui me tient à coeur, ce sont les déplacements du quotidien. Être à l'écart des métropoles ou des grands axes de communication, c'est insupportable. Mais je pense également à toutes les personnes qui n'ont pas d'autre option que leur véhicule individuel pour se déplacer, à ceux qui n'ont pas de voiture ou qui ne peuvent pas conduire. Le développement des infrastructures peut être nécessaire, mais il n'est pas forcément suffisant. Je suis convaincue que l'on ne réglera pas les problèmes des territoires sans proposer des alternatives à l'usage individuel systématique de la voiture. Outre la question de l'enclavement, c'est aussi celle du pouvoir d'achat et de la capacité pour tous à accéder aux emplois, à la formation et aux services, ainsi que les enjeux de la protection de notre environnement, qui sont posés. posés. Pour lutter contre les fractures territoriales, sociales, environnementales, il faut une vision globale de la mobilité. C'est bien toute la philosophie du projet de loi d'orientation des mobilités, qui, outre la programmation des infrastructures, a pour ambition d'apporter de vrais outils pour permettre aux territoires de proposer des solutions concrètes. Cela passe notamment par une amélioration de la gouvernance, mais aussi par l'innovation, qui, j'en suis convaincue, offre une grande diversité de solutions adaptables aux territoires. Tout l'enjeu est que ces innovations puissent se déployer grâce à la prise de compétence mobilité sur tout le territoire. L'État accompagnera les territoires dans leur démarche. C'est d'ailleurs tout l'objet de la démarche France Mobilités, lancée à la suite des assises. Nous avons choisi d'accompagner les territoires sans attendre la loi, pour faire ce qui est déjà possible et anticiper ce qui le sera demain. Plus de cinquante territoires, essentiellement ruraux, ont déjà été sélectionnés pour leur démarche. Les projets retenus sont divers et illustrent parfaitement la créativité et l'ingéniosité sur nos territoires. Que ce soient des expérimentations d'autopartage en milieu rural, des véhicules autonomes dans des territoires peu denses, des projets visant à structurer l'offre de mobilité en milieu rural, ce sont autant de réponses possibles aux problèmes de mobilité du quotidien de nos concitoyens. Aussi, en conclusion, je ne puis que partager les constats et les grands enjeux portés par cette proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c'est un rural, un montagnard qui vous parle, au nom des territoires. Ruraux et montagnards, nous savons ce que c'est l'enclavement. C'est un quotidien qui crée un sentiment d'éloignement, une réalité d'éloignement quand le monde bouge autour de vous, mais que vous ne possédez pas les moyens de vous connecter, donc de faire bouger votre quotidien, d'être dans le, comme on dirait dans la ... Désenclaver nos zones rurales est vital pour notre développement. Les maîtres mots ici ne sont-ils pas l'accessibilité, la mobilité et la connexion ? La proposition de loi dont nous discutons rappelle les difficiles vérités des territoires enclavés, aggravées par la loi portant nouvelle sentiment d'abandon, fractures économiques et sociales, creusement des inégalités. Il est grand temps d'agir. Cette proposition de loi n'est que l'ébauche d'un réel plan attendu par nos territoires. Ceux-ci ont besoin d'un véritable plan Marshall, avec des perspectives à long terme concernant la politique des transports.

Si cette proposition est donc l'ébauche, nous pourrions nous attendre à ce que le projet de loi d'orientation des mobilités soit le plan Marshall pour nos transports. Vous affirmiez à ce sujet, madame la ministre, lors de votre audition au Sénat la semaine dernière, que le dès la campagne électorale et le début de son mandat, avait souhaité faire une pause dans les grands projets, afin de prendre le temps de construire une rupture, avec un objectif majeur : répondre aux besoins de tous et dans tous nos territoires. Nous voilà avec un projet de loi d'orientation doté d'un objectif qui laisse circonspect. Nous ne vous demandons pas de « construire une rupture », mais de construire des routes sûres, d'améliorer les dessertes ferroviaires et d'accélérer le numérique dans tous les territoires

Sa réalisation serait un réel signe de considération pour nos territoires ruraux et enclavés. Paris-Clermont en deux heures trente, et des ruraux à moins de soixante minutes d'automobile d'une gare desservie par une ligne à grande vitesse, voilà du concret contre le désenclavement

Il y a ici un réel sujet d'actualité avec la redéfinition actuelle des lignes d'Air France et de HOP !. Le Puy-de-Dôme peut vous en parler ! Le « transport virtuel » est aussi essentiel- je veux parler de la couverture numérique.

Aujourd'hui, les Français parcourent en moyenne 45 kilomètres par jour, contre 5 kilomètres dans les années soixante. La distance moyenne entre le lieu de résidence et le lieu de travail est de 28 kilomètres pour un habitant des zones rurales, et la distance moyenne du domicile aux commerces a augmenté de 30 % en quinze On ne peut donc que corroborer la nécessité de ne pas adopter des normes centralisées qui s'imposent sans distinction, comme cela a été fait pour les 80 kilomètres par heure. Donner la compétence aux présidents de département et aux préfets de relever la vitesse maximale autorisée sur les routes dont ils ont la gestion est positif, car les réalités du terrain seront prises en compte. Toutefois, permettre de relever la vitesse ne doit pas aboutir à mettre en cause la responsabilité de nos élus face à une mortalité qui continuera sur nos routes, si faible soit-elle.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comment améliorer les déplacements dans les zones rurales et périurbaines ? Comment garantir à chacun la possibilité de se déplacer pour accéder à l'emploi, à la formation, à la santé, à la culture ? En somme, comment désenclaver nos territoires ? Ces questions fondamentales ont fait l'objet, vous l'avez dit, madame la ministre, de débats riches et intenses à l'occasion des Assises nationales de la mobilité. En effet, nous le savons, nos concitoyens ne sont pas égaux face aux transports. Parmi les formes d'inégalité qui limitent la mobilité, le facteur géographique d'éloignement dans les territoires de faible densité est une réalité qui touche tous nos concitoyens. Ainsi, les territoires moins denses, ruraux, périurbains, les petites villes et villes moyennes, les quartiers périphériques peuvent être fragilisés au regard d'une mobilité qui est loin d'être aisée. Cette fragilité, cette fracture, cet enclavement sont vécus au quotidien par des millions de nos concitoyens. Or l'accès quotidien à l'emploi, à l'éducation, à la santé, aux commerces, aux relations sociales, aux loisirs est une condition essentielle d'exercice des droits fondamentaux de liberté, d'égalité et de citoyenneté, et c'est à ce titre que le désenclavement des territoires doit être une priorité. Dans son rapport, notre collègue Jean-Pierre Corbisez nous rappelle que la France compte de nombreux territoires enclavés. Cette situation pose des problèmes quotidiens à nos concitoyens, qui rencontrent des difficultés à accéder à un emploi, à des services publics ou à des biens de consommation courants. La persistance de cet enclavement se double d'une montée des inégalités économiques et sociales entre les territoires et alimente un sentiment d'éloignement d'une partie de la population. Ce sentiment d'abandon d'une certaine frange de la population s'est cristallisé, ces derniers mois, autour du mouvement des gilets jaunes. En réponse, le Président de la République a engagé un grand débat national permettant à tout un chacun de faire valoir son opinion. Ce grand débat est en cours et il serait opportun d'en attendre l'issue pour proposer les solutions les plus adéquates, en matière de désenclavement comme pour d'autres questions essentielles. L'enclavement des territoires résulte avant tout d'une offre de mobilité, notamment en transports collectifs, insuffisante, ainsi que d'un manque d'infrastructures de transport adaptées, et chacun peut constater aujourd'hui à quel point cette absence de solution de mobilité alimente un sentiment d'abandon d'une partie de notre population. Concernant l'aérien, point saillant du texte, bien que les élus locaux perçoivent le plus souvent la force symbolique de la présence d'un aéroport sur leur territoire, le rapport du Commissariat général à l'égalité des territoires, le CGET, de janvier 2017 insiste sur la nécessité d'études approfondies sur les recouvrements de zones d'attraction des aéroports, avant d'examiner localement une offre aéroportuaire. Le transport aérien contribue-t-il pertinemment au désenclavement des territoires les moins desservis en France métropolitaine ? Le prix moyen du billet pour les petites lignes aériennes pose la question d'une véritable perspective de désenclavement de ces territoires. En effet, le coût du transport qui permettra le désenclavement de ces territoires aura une influence sur le nombre de citoyens touchés par la mesure. Or on peut facilement douter que le coût du transport aérien permette un désenclavement le plus large possible pour ces territoires. Le montant de subventions que nécessiterait un tel programme est à comparer au bénéfice qu'en retirerait l'ensemble des populations de ces territoires. Aussi, il me semble que certaines mesures de cette proposition de loi, notamment celles relatives à l'aérien, mériteraient d'être creusées et nécessiteraient une étude d'impact approfondie, en particulier sur le plan financier. Avant de légiférer, il conviendrait d'anticiper le montant des subventions qui seraient nécessaires au développement d'aéroports de désenclavement. Oui, nous voulons tous contribuer au désenclavement des territoires. Le métropolitain que je suis peut vous dire que le désenclavement est également nécessaire sur certaines parties géographiques des métropoles. Pour autant, cette proposition de loi arrive un peu tôt, puisqu'il serait opportun que nous attendions les conclusions du grand débat national et elle intègre bien des points que nous examinerons à partir du 19 mars prochain dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Si l'on ne peut qu'être favorable au désenclavement des territoires, je le disais, la question du financement reste posée. À L'heure où les trois quarts de nos concitoyens utilisent leur voiture pour leurs trajets domicile-travail, la loi d'orientation des mobilités propose d'apporter des solutions de substitution à l'usage individuel de la voiture, ce qui semble un tantinet dissonant avec l'objet de cette proposition de loi. Dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, l'accent est mis sur le travail avec les collectivités locales, qui permettra de bâtir des réponses au désenclavement à partir des réalités du terrain. Avec une méthode claire, vous l'avez rappelé, madame la ministre, le Gouvernement doit s'engager sur des projets qu'il sait pouvoir réaliser et qui répondent aux besoins des habitants, en s'assurant de l'effectivité des ressources par rapport aux engagements pris. J'ai déjà pu constater l'efficacité de la méthode lors de la signature du contrat de transition écologique du territoire de la Sambre-Avesnois, dans le cadre duquel la mise à 2x2 voies de la RN 2 a été annoncée, avec les financements afférents, après plus de quarante ans d'attente. De la même manière, je voudrais ici rappeler le pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, lancé sur l'initiative du ministre Mézard, doté d'une enveloppe de 5 milliards d'euros, qui reconnaît et consolide les villes moyennes dans leurs fonctions de centralité, car elles irriguent les communes petites et rurales environnantes, qu'il s'agisse de l'offre de santé, d'éducation, d'accès au ferroviaire, au commerce, à l'emploi ou aux services administratifs. En définitive, le désenclavement des territoires doit être une préoccupation majeure, particulièrement dans notre assemblée. Néanmoins, nous sommes à l'aube du démarrage de la discussion sur la loi d'orientation des mobilités. Même si ce texte soulève de vraies questions, qui convergent avec l'ambition du Gouvernement, je pense que celles-ci pourront largement être débattues et traitées dans le cadre de l'examen et de l'enrichissement de la loi d'orientation des mobilités. C'est pourquoi le groupe La République En Marche s'abstiendra. La

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi proposée par le groupe du RDSE visant à faciliter le désenclavement des territoires. Il est évident que nous partageons le constat initial de ce texte, lorsqu'il pointe l'accroissement de la fracture territoriale et l'enclavement de certains territoires ruraux confrontés à un manque d'attractivité et à une disparition des services publics. La mobilisation depuis des mois des gilets jaunes, exaspérés notamment par l'injustice territoriale, témoigne de cette paupérisation qui frappe les zones périurbaines, les villes petites et moyennes. Ils voient leurs commerces disparaître les uns après les autres, la vacance grandissante des logements qui ne trouvent pas de locataires et l'accessibilité aux services publics locaux se réduire comme peau de chagrin. Tout cela nourrit un sentiment très fort d'abandon des pouvoirs publics. Face à l'expression d'un tel attachement à l'égalité des territoires, on en viendrait presque à se demander pourquoi notre éminent collègue a participé à un gouvernement qui, par ses mesures, a, pas à pas, aggravé la fracture territoriale effet, et c'est le moins que l'on puisse dire, le bilan du Gouvernement en la matière n'est pas bon. La réforme ferroviaire va immanquablement conduire à l'abandon d'un certain nombre de lignes du quotidien jugées trop peu rentables. La réforme de la justice menace les petites juridictions. Sans attendre la réforme de la santé, l'accès aux soins se réduit. On pense notamment aux maternités qui ferment les unes après les autres. Pis encore, l'épée de Damoclès de la suppression de 70 000 fonctionnaires territoriaux pèse sur les collectivités locales. À la lumière des enjeux évoqués, à quelques jours du débat sur la loi d'orientation des mobilités, vous comprendrez dès lors qu'au-delà de son objectif ambitieux, le contenu de cette proposition, notamment dans sa version initiale, nous a semblé à la fois lacunaire et totalement inadapté. lacunaire, car les solutions contre l'enclavement se limitent au prisme de l'accessibilité physique des territoires. S'il s'agit évidemment d'un des éléments de l'enclavement, celle-ci n'est ni exclusif ni suffisant. Bien sûr, ces territoires souffrent de l'absence de transports, et surtout d'ailleurs de solutions de mobilités internes. Cependant, si de nombreux Français se relaient sur les ronds-points tous les samedis depuis des mois, c'est aussi parce qu'ils souffrent durement de la fermeture des écoles, des hôpitaux, des bureaux de poste et autres maternités. Aucune mention n'est faite dans ce texte des impacts de la mise en concurrence des territoires, des politiques de réduction de la dépense publique ou de celles qui ont conduit à libéraliser les services publics et à réduire leur présence territoriale par la privatisation. Les services publics sont pourtant essentiels pour résorber la facture territoriale.

inadapté, car l'égalité territoriale ne se résume pas à relier des zones-dortoirs à des métropoles qui concentreraient tous les services. Ce n'est pas notre vision de l'aménagement du territoire. Ce prisme est tellement réducteur que l'on en viendrait presque à se demander si cette proposition de loi a un autre objet que de faciliter la vie de quelques responsables politiques et acteurs économiques qui font des allers et retours fréquents vers la capitale ou les métropoles régionales ... Alors que la question climatique se pose avec une acuité toute particulière, comment peut-on, comme cette proposition de loi, n'envisager la mobilité que par les airs et par la route en omettant le rail ? Construire des aéroports tous les 200 kilomètres est une vision de l'aménagement du territoire des années soixante-dix, que n'aurait d'ailleurs pas renié Pompidou. De cette époque, nous avons hérité d'une soixantaine d'aéroports peu utiles et déficitaires, que l'on maintient sous perfusion d'argent public, quand on laisse mourir les lignes de chemin de fer. Dans l'Isère, que je connais bien, le département vient de voter une subvention de plus de deux millions d'euros pour maintenir à flot l'aéroport de Grenoble-Alpes-Isère. A-t-on vraiment envie de flécher les dépenses publiques vers un mode de transport aussi peu rentable qu'écologiquement polluant ? Par ailleurs, avec quel argent comptez-vous le faire ? Pas l'ombre d'une piste de financement n'est avancée dans la proposition de loi. La fracture territoriale ne se résorbera pas par le simple amas de bonnes volontés et par des textes de loi inapplicables, mais avec des moyens concrets. Elle implique de revitaliser les territoires par la création d'emplois ; par une véritable politique de soutien à l'agriculture, à l'artisanat, par une reconquête industrielle et par la relocalisation des sites de production. Penser l'aménagement du territoire nécessite d'inscrire au coeur des politiques de mobilité les enjeux de report modal de la route vers le rail, et il nous semble incroyable qu'il n'en ait pas été fait mention une seule fois dans ce premier jet de proposition de loi. Car ce sont les lignes de chemin de fer régionales qui repeuplent les campagnes, pas les autoroutes, qui les traversent comme des tunnels, ou les aéroports. Nous saluons néanmoins les évolutions positives du texte en commission, et je tiens ici à remercier notre rapporteur et notre collègue Ronan Dantec, dont les amendements remplacer le critère de distance avec un aéroport par celui de la proximité avec une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Ce changement fait sens. Il en va de même pour la réécriture de l'article 2, qui était flou et qui laissait penser que l'État pourrait déroger aux normes environnementales de construction des infrastructures dans certains territoires enclavés, ce qui ne pouvait constituer une solution acceptable. Néanmoins, cela ne suffira pas pour voter en faveur d'un texte qui propose une vision aussi réductrice d'un enjeu aussi majeur. Nous choisissons donc de nous abstenir. La

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi aborde un objectif auquel nous ne pouvons qu'adhérer : le nécessaire désenclavement des territoires, pour trouver une réponse aux fractures territoriales, sociales et démographiques qui traversent notre pays. Il faut en effet résolument s'attaquer aux causes de l'enclavement et lutter contre un sentiment qui se généralise aujourd'hui, celui de l'exclusion d'une grande partie de nos concitoyens. Cohésion des territoires et lutte contre la marginalisation vont de pair. À ce titre, nous soulignons la qualité du travail du rapporteur et de la commission, qui a permis d'améliorer le texte sur plusieurs points, notamment sur l'objectif de désenclavement à l'horizon 2025, dont devront tenir compte les schémas nationaux des infrastructures de transports et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Nous soutiendrons donc ce texte. 26 % du territoire national accueillent 5,6 % de la population. Ces territoires se distinguent par une faible densité, bien sûr, souvent de faibles ressources économiques, un départ des forces vives et des jeunes et le vieillissement de la population. Si cette situation est devenue critique dans les territoires les plus enclavés, elle est le fruit de notre histoire, de la métropolisation et d'une décentralisation qui n'a pas complètement joué son rôle. Les dynamiques urbaines de la France ont concentré mécaniquement l'activité économique porteuse d'emplois, les métiers qualifiés ou d'avenir et la création de richesses. Il en découle un sentiment diffus de malaise dans les campagnes, renforcé par l'isolement géographique. Cette « France périphérique » ne compte plus les maternités et les classes qui ferment, ni les lignes de trains supprimées. Elle subit aussi la désertification médicale. Dans l'ensemble de ces territoires, le nombre de communes équipées en services publics a fortement diminué depuis les années quatre-vingt. La part des gares ferroviaires y a, par exemple, baissé de 41,8 %. Pour elles, l'enjeu du désenclavement est essentiel. Seulement 14 % des 15-29 ans vivent dans l'espace rural. Il faut donc faire émerger les projets ruraux, car ces territoires sont un vivier futur : ils regorgent d'espaces économiques actifs, mais aussi d'une qualité de vie indéniable. La ruralité doit prendre sa part entière aux défis d'aujourd'hui : la transition énergétique, le numérique, la mobilité. La proposition de loi n'évoque pas le devenir des petites lignes, pourtant indispensables dans le report modal, le mix des transports. Seraient-elles d'ores et déjà condamnées ? Madame la ministre, vous avez récemment affirmé que l'entretien des réseaux avait été négligé et qu'il fallait réinjecter des finances pour « s'occuper de la mobilité et des déplacements du quotidien. Ce que nous regrettons, une fois de plus, ce sont les chiffres. Depuis 2011, quelque 744 kilomètres de petites lignes ont été fermés et la loi pour un nouveau pacte ferroviaire ne laisse rien présager de bon. Plusieurs syndicats ont déjà dénoncé « le sabotage des projets de maintien des petites lignes de la part de SNCF Réseau Dans ma région, l'Occitanie, ce sont 40 % des petites lignes qui fermeraient à l'échéance 2021. Vous annoncez vouloir favoriser le développement des véhicules électriques pour sortir de la dépendance au pétrole, mais la mobilité de demain exige également la restauration et le maintien de ces petites lignes. Restructurer les réseaux en tenant compte de l'objectif de désenclavement est incontournable. Il faut renforcer les pôles d'échanges autour des lignes existantes. On supprime les très petites lignes, mais parfois aucune autre infrastructure n'existe. C'est le volontarisme politique qui valorisera nos territoires ruraux et donnera du sens à la mobilité sociale et professionnelle. L'enclavement géographique ne peut plus avoir pour corolaire le déficit des services publics, la marginalisation numérique et la persistance d'infrastructures de transports insuffisantes. Quels que soient les efforts de ces territoires pour s'en sortir, les initiatives seront en partie entravées. Ces territoires sont logiquement aujourd'hui le royaume de la voiture individuelle, dont il est nécessaire de sortir, nous sommes d'accord. Ainsi, quelque 80 % des personnes travaillant dans une commune où elles ne résident pas utilisent leur véhicule. L'Insee révèle que 58 % des actifs qui travaillent à moins d'un kilomètre de leur lieu de travail s'y rendent en voiture. Les véhicules électriques pour sortir de cette dépendance au pétrole doivent s'accompagner d'une réelle politique en faveur du ferroviaire. Nous espérons que vous en tiendrez compte dans la loi à venir sur les mobilités. Qui dit mobilité dit, enfin, vitesse abaissée à 80 kilomètres par heure. Appliquée depuis le 1 juillet 2018 sur les routes secondaires et très critiquée par bon nombre d'élus locaux et de « gilets jaunes »- c'est l'actualité -, cette mesure illustre une prise de décision unilatérale, qui n'a pas su tenir compte, notamment, des préconisations sénatoriales. Le groupe de travail du Sénat avait pourtant relevé les insuffisances de l'expérimentation conduite. Il avait souligné la nécessité de revoir la méthode envisagée par le Gouvernement, au bénéfice d'une réduction de la vitesse sur les routes les plus accidentogènes, en incluant un travail avec les départements.

Cela fait mal aux tripes », m'a-t-il confié. Et de conclure : « La ruralité est en train de mourir ». Il s'agit là non pas de nostalgie, mais d'un constat amer, d'une inquiétude, d'un profond désarroi. Cette proposition de loi, madame la ministre, doit vous inviter à l'attention et à la vigilance, car nous ne pouvons laisser mourir nos campagnes. Le dépeuplement et la friche guettent un certain nombre de territoires hyper-ruraux et vieillissants. Les métropoles peuvent-elles continuer à croître et à se densifier sans fin ? Oui ! N'avons-nous plus besoin des paysans ? Le développement durable n'est-il pas lié à la proximité ? Le changement climatique, les problèmes de pollution, les enjeux de santé alimentaire, tout concourt à agir pour un développement durable qui ait du sens, c'est-à-dire qui s'envisage dans la proximité et replace nos territoires enclavés au coeur des préoccupations qui doivent être les vôtres, afin que ceux-ci ne deviennent pas les territoires oubliés, voire perdus de la République. La France est vivante de ses campagnes, de son riche patrimoine, de ses terroirs gourmands, de ses paysages façonnés par les paysans, du foisonnement des petites routes qui irriguent un territoire national apprécié du monde entier. Ne sommes-nous pas le pays le plus visité au monde ? Gouverner, c'est être visionnaire, c'est se laisser traverser par tout ce que le pays murmure, c'est s'imprégner et transcender, c'est anticiper et préparer l'avenir pour être utile au pays. La parole

les collectivités territoriales ont été amenées à payer une quote-part financière. C'est exact ! La SNCF s'était engagée, en échange, à offrir une desserte cadencée

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous procédons aujourd'hui à l'examen d'une proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires. De toute évidence, nous partageons tous le même diagnostic et les mêmes objectifs, à savoir agir sur les causes de l'enclavement en améliorant la qualité et l'accessibilité des moyens de transport dans les zones les plus reculées du territoire métropolitain. Il est en revanche étonnant, pour ne pas dire dérangeant, d'avoir à débattre de thématiques qui seront au coeur de nos échanges en commission dans moins de deux semaines, lorsque nous examinerons le projet de loi d'orientation des mobilités. Les nouvelles formes de gouvernance territoriale, la capacité offerte à chaque territoire de créer des solutions sur-mesure, l'organisation multimodale et intermodale, la programmation des grandes infrastructures de transport sont autant de réponses que la LOM devra apporter pour que chaque zone blanche actuelle ne le soit plus demain, dans un réel souci d'aménagement du territoire. N'oublions pas non plus que la question du financement, par l'État et les collectivités locales, reste entière. Elle devra être résolue. Nous pouvons donc nous interroger sur le choix d'étudier aujourd'hui cette proposition de loi. Un débat sur le sujet aurait à mon sens était plus pertinent. Mais puisque nous avons choisi de faire un échauffement, lançons-nous, mes chers collègues La lecture attentive de vos propositions m'amène à formuler quatre remarques. En premier lieu, nous pourrions nous pencher sur l'empilement de lois, de structures et de documents de programmation : LOADT, LOADDT, SRU, DTA, SCOT, PDU, SNIT, SRADDET, PLU, et j'en oublie sûrement Alors que la situation actuelle nous amène à nous interroger sur l'état de nos finances publiques et sur l'efficience de nos administrations, nous avons un bel exemple de ce que la technostructure et le millefeuille administratif sont en capacité de produire en complexité, en schémas directeurs rarement cohérents et le plus souvent réalisés selon des temporalités différentes. De surcroît, comme l'a récemment souligné M. Didier Migaud dans notre hémicycle,

Dresser un inventaire à la Prévert est aisé et pourrait faire miroiter à nos concitoyens l'arrivée d'équipements qui ne peuvent être financés ou dont la réalisation mobiliserait des sommes déraisonnables.

Impliquée depuis plus de vingt ans sur la thématique des mobilités, je ne compte plus le nombre de promesses non tenues, le nombre d'études réalisées et de projets absurdes achevés en opposition à toutes les programmations, aussi brillantes En tant que membre du Conseil national de la transition écologique, j'aimerais que nous nous interrogions également, mes chers collègues, sur la pertinence écologique de nos propositions. Bien sûr, chaque cas est à étudier de façon spécifique, l'avion pouvant être parfois la seule solution. Mais ne nous interdisons pas de revoir nos certitudes un car doté des dernières technologies antipollution est une alternative crédible pour remplacer une petite ligne ferroviaire propulsée par une machine thermique d'un autre temps. Enfin, en tant que corapporteur, avec mes excellents

pour que les limitations de vitesse soient définies localement, en fonction de la dangerosité effective des voies, sans omettre la vitesse des poids lourds ni la qualité des chaussées. Il me semble que les récentes déclarations du chef de l'État et du Premier ministre prouvent que nous avons été entendus, bien aidés, je vous le concède, par une pression populaire sans précédent, qui parfois est justifiée- en l'occurrence, elle l'était. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, sans vouloir mettre à mal le travail réalisé par le groupe du RDSE, il me semble opportun de prendre rendez-vous le 19 mars prochain dans ce même hémicycle,

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

Pourtant, l'enclavement de certains de nos territoires reste une réalité, qui vient fracturer la cohésion sociale, accroître les disparités économiques et renforcer le sentiment d'exclusion. Nous le savons, le réseau routier joue un rôle fondamental dans les zones rurales, que soit pour leur développement économique et touristique, pour l'implantation d'entreprises, pour faciliter l'installation de retraités ou de jeunes actifs, mais aussi le développement de transports collectifs performants. Et c'est sans compter sur les décisions prises sans aucune considération des territoires, comme le montre encore l'exemple récent de la mobilisation des élus des Hauts-de-France pour le maintien des dessertes régionales des TGV. Le désenclavement des territoires doit être l'un des objectifs prioritaires, avec la mise en place d'une stratégie globale regroupant la programmation des investissements relatifs aux infrastructures de transport, l'entretien des routes existantes, la mise en place de réseaux ferroviaires et aériens performants et accessibles, le développement des transports collectifs, ou encore de solutions de rechange, comme le télétravail. En outre, pour bien pour bien en traiter les causes, il faut d'abord en livrer une définition précise et objective, ce qui, comme le montrent de nombreux rapports passés, est loin d'être évident. pourtant indispensable pour définir les objectifs d'une politique pertinente et guider de façon éclairée les choix de la puissance publique. On peut ainsi s'interroger sur la pertinence de la norme des 45 minutes et 50 kilomètres pour décrire les situations d'enclavement vécues au quotidien par les habitants de certains territoires. La question du temps passé chaque jour dans les transports peut aussi être une façon de traduire au mieux ce sentiment au quotidien. Surtout en Île-de-France ! Il n'est donc pas évident de définir un critère objectif pertinent, c'est-à-dire le type d'isolement qui pose réellement des problèmes au territoire concerné. Cette notion est aussi étroitement liée à notre vision très centralisée des territoires. Et il est important, également, de prendre en compte la perception des habitants pour définir une zone enclavée. Ainsi, un citoyen peut se sentir isolé, non pas parce qu'il se trouve loin d'une ville ou d'un gros centre-bourg, mais parce qu'il est dans une zone blanche non couverte par le numérique. naturellement à prendre en compte dans les politiques mises en place. Les infrastructures de transport doivent nécessairement prendre en compte la stratégie locale pour permettre une bonne articulation de l'infrastructure nouvelle avec l'ensemble du système de transport existant et ainsi assurer, autour d'un véritable projet, le développement optimal des territoires. Je soutiens également la position de la commission sur la réglementation de la vitesse sur les routes. La réduction de la vitesse maximale autorisée à 80 kilomètres par heure sur les routes secondaires a été mal vécue

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, avec cette proposition de loi, le groupe du RDSE réaffirme l'attachement qu'il porte et qu'il a toujours porté à la ruralité et aux territoires fragiles. Aussi, je tenais à remercier Jacques Mézard de cette belle initiative. On parle depuis longtemps de « diagonale du vide », de « France périphérique » et de territoires enclavés. Derrière ces expressions, se cache une seule et même réalité : l'éloignement. L'éloignement de l'emploi, même avec tous les soutiens possibles, comme le tout récent programme du Gouvernement « territoires d'industries », car, sans désenclavement, il n'y a pas d'attractivité économique. L'éloignement des formations supérieures, qui font que claque année de trop nombreux jeunes quittent nos territoires ruraux pour aller travailler ou étudier dans les métropoles. L'éloignement des spécialistes de santé, qui nous plonge dans une précarité médicale, avec des fermetures de services toujours plus grandes et des alternatives toujours plus rares. Parler d'enclavement, enfin, c'est parler de manière plus générale de l'éloignement de l'ensemble de nos services publics, bureaux de poste, trésoreries et écoles. C'est aujourd'hui une réalité insupportable. Le préalable à cet éloignement est l'accès aux infrastructures routières, ferroviaires et aériennes, comme l'a rappelé mon collègue Jean-Yves Roux. Cette proposition de loi, nous en sommes bien conscients, ne viendra pas révolutionner les problèmes énoncés, mais elle pose une première pierre et devrait permettre d'amorcer un travail bien plus global, qui, nous l'espérons, trouvera aussi des débouchés dans la prochaine loi d'orientation des mobilités. La première réponse à apporter est l'investissement dans nos infrastructures de transport pour sortir ces territoires de l'isolement.

À ce titre, nous soutiendrons un amendement visant également à prendre en compte la distance aux préfectures et sous-préfectures, clin d'oeil symbolique, mais ô combien d'actualité, à l'idée qui prévalait lors de leur création, celles-ci devant être situées à moins d'une journée de cheval des communes.

en permettant la réalisation d'infrastructures plus légères et moins coûteuses, dans un contexte budgétaire toujours plus restreint et avec des collectivités qui doivent jongler avec la contractualisation.

Ainsi, mon territoire, comme de nombreux autres, a investi dans les liaisons internes afin de garder son attractivité, pour les entreprises comme pour les ménages. Si, actuellement, l'État et la région sont compétents pour organiser les liaisons d'aménagement du territoire, les autres collectivités, à l'image des départements et des EPCI à fiscalité propre, peuvent intervenir dans le financement de ces lignes soumises à une obligation de service public. En fait, elles n'ont pas d'autres choix, si elles souhaitent conserver un accès rapide aux grands centres de décision. L'objectif de l'article 3 est de réaffirmer cette possibilité, mais les membres de mon groupe auraient souhaité aller plus loin, en laissant l'initiative de l'organisation de ces liaisons d'aménagement aux aux collectivités du territoire, sans autorisation obligatoire préalable de l'État. Si ces liaisons sont vitales pour nos territoires et qu'elles sont aussi une vraie réussite, leur gestion laisse parfois les élus financeurs dubitatifs, tant sur le fonctionnement que sur les résultats d'exploitation de ces lignes. N'oublions pas, en effet, le contexte financier pour les collectivités, contraintes par l'État de ne pas augmenter leurs dépenses de plus de 1,2 %, selon les directives actuelles. Si je prends l'exemple de la ligne Tarbes-Orly, nous sommes sur un taux de remplissage avoisinant les 80 avec une croissance du nombre de passagers de plus de 4 % l'année dernière. Malgré cela, on nous explique que cette ligne est déficitaire et que, pour la maintenir, le conseil régional, le conseil départemental et l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées doivent payer.

permettant un plus large contrôle de l'État sur ces lignes soumises à une obligation de service public. L'État doit s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur maintien. Pour les collectivités qui les financent en large partie, il est fondamental de savoir où va l'argent investi sur leurs frais de fonctionnement, notamment s'il est bien investi.

Sur ce sujet, la question n'est pas d'être pour ou contre cet abaissement- le débat est d'ailleurs large dans mon groupe. Il s'agit de faire confiance aux élus locaux, qui connaissent leurs territoires. pour combattre cet éloignement qui organise depuis de trop nombreuses années les inégalités dans nos territoires, il serait nécessaire d'établir une véritable équité territoriale. Mon groupe, vous l'aurez compris, mes chers collègues, votera cette proposition de loi issue de ses rangs. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la présente proposition de loi vise à agir directement sur les causes de l'enclavement des territoires, en améliorant la qualité et l'accessibilité des moyens de transport dans ces zones. Cette problématique a une résonnance particulière pour le territoire montagnard que j'ai l'honneur de représenter. En effet, si la montagne est un lieu d'exception pour tous les Français, c'est surtout et avant tout un espace singulier où des habitants vivent et travaillent toute l'année des zones où les trajets ne se traduisent pas en kilomètres, mais en temps de parcours ; des territoires riches de leurs activités saisonnières, mais aussi artisanales, agricoles, forestières et industrielles ; des territoires qui connaissent également des difficultés liées à l'enclavement ou à des enjeux environnementaux majeurs des territoires, enfin, dont l'avenir est fragilisé par le réchauffement climatique. En montagne plus qu'ailleurs, les actes de la vie courante peuvent souvent s'avérer compliqués, voire impossibles l'hiver, avec de nombreux cols fermés et parfois des accidents naturels coupant les voies d'accès. Cet état a même été reconnu par le traité de Lisbonne, adopté en 2009, qui range la montagne parmi les « régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents » et devant bénéficier d'une priorité en matière de politique de cohésion économique et sociale. Pour faire vivre la promesse d'égalité entre les territoires, le premier enjeu concret pour chacun, c'est l'accès et la liberté de se mouvoir. Face aux changements climatiques et aux évolutions de la société, les habitants de la montagne doivent être rassurés sur la pérennité de leur mode de vie. Or, les réalités de nos territoires semblent depuis longtemps avoir été oubliées dans l'élaboration des politiques publiques menées successivement depuis de nombreuses années. Comment ne pas évoquer ici l'impérieuse nécessité de désenclavement du Chablais, en gestation depuis de très nombreuses années ? Cette région, qui s'étend sur 900 kilomètres carrés et recense environ 100 000 habitants, connaît une forte activité, qui lui impose de modifier son mode d'aménagement. Chaque jour, ce sont plus de 20 000 actifs qui quittent le Chablais pour se rendre à leur travail, en France métropolitaine, mais aussi en Suisse, avec un taux de sortie qui frôle les 34 %. L'utilisation du véhicule personnel prédomine pour huit actifs sur dix, faute, à ce jour, d'un mode de transport en commun adéquat. Aussi, je profite de cette intervention pour soutenir avec force le projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et Thonon-les-Bains, dernier barreau manquant de l'axe routier structurant devant relier l'A 40 à Thonon. Ce projet, porté par l'État, constitue une priorité absolue pour ce territoire. Je ne saurais également passer sous silence l'urgence de la modernisation du réseau ferroviaire, préalable indispensable à la mise en oeuvre d'une mobilité douce, cadencée et capable d'être compétitive par rapport à la voiture. Si l'arrivée prochaine du Léman Express offrira un service de qualité à la zone frontalière, nous attendons une amélioration rapide du réseau ferroviaire et du cadencement en direction d'Annecy, Évian et Chamonix. Enfin, puisque l'article 2 de ce texte vise à faciliter la construction d'infrastructures moins lourdes dans les zones enclavées, il conviendra de favoriser l'émergence de projets d'ascenseurs de vallée, au moyen d'un cadre juridique plus performant. Le développement du transport par câbles constitue une alternative crédible et pertinente au transport routier, notamment en montagne. Cette solution est particulièrement adaptée au franchissement de dénivelés et d'obstacles naturels, sans émission de polluants atmosphériques, d'autant plus que la France possède une longue tradition d'ingénierie en la matière, ainsi que l'un des leaders mondiaux dans ce domaine. Telles sont, mes chers collègues, les attentes de la montagne s'agissant de cette proposition de loi, que je soutiendrai sans réserve, en espérant que, plus qu'à des paroles, ce texte donnera lieu à des actes et à des engagements forts en faveur de la mobilité dans nos territoires. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la première manière de désenclaver un territoire, c'est d'assurer son raccordement aux autres espaces territoriaux. Au regard du poids économique de Paris et de la région Île-de-France, l'une des conditions du désenclavement est aussi de relier nos territoires à Paris. Les usagers le mesurent quotidiennement de Metz vers Paris, tout comme les travailleurs frontaliers qui, chaque matin, affrontent un véritable calvaire sur les lignes TER vers Luxembourg. Vous comprendrez donc, madame la ministre, mes interrogations récentes décisions de la SNCF de supprimer des TGV sans aucune annonce officielle préalable, le tout dans une attitude d'opacité qui ne peut que susciter interrogations et mécontentements. À l'heure des réseaux sociaux, pourtant largement utilisés par la SNCF, cette dernière ne communique plus. Elle n'a, par exemple, pas jugé utile de communiquer sur la disparition de certains TGV vers ou au retour de Paris au début du mois de décembre, allant même jusqu'à mentir sur ce

P-DG de la SNCF semble lui-même peu soucieux de répondre à ceux, notamment les parlementaires, qui le questionnent, nos courriers d'octobre 2018 étant toujours sans réponse.

La SNCF agit unilatéralement et autoritairement sur tous les sujets. Pourtant, nos collectivités sont mobilisées et demandent toutes à être parties prenantes, aux côtés des associations d'usagers, d'un véritable débat des mobilités dans nos territoires : débat sur la LGV, mais aussi sur toutes les autres lignes de l'axe Nancy-Luxembourg et sur le désenclavement des espaces de l'Est mosellan ou des bassins de vie frontaliers de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne. Je vais illustrer mon propos par l'exemple de la suppression sans concertation de la ligne entre Saint-Dié et Épinal, qui contraint les habitants de deux aires urbaines de 50 000 et 100 000 habitants à ne se déplacer qu'en voiture ... Quel progrès pour l'environnement ! ! Des exemples de ce type, chacune et chacun de mes collègues ici présents en a un en tête. À l'heure du grand débat, mais surtout des mouvements sociaux de ces derniers mois, le silence de la SNCF est d'autant plus absurde et incompréhensible. Comment désenclaver nos territoires si le premier service public de mobilité n'est plus assuré ? Comment désenclaver nos territoires si la concertation est impossible ? Autant de questions sur lesquelles les citoyens de nos territoires attendent la SNCF, mais vous attendent aussi, madame la ministre.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je remercie tout d'abord nos collègues d'avoir porté devant notre assemblée le sujet de l'enclavement des territoires. une réalité qui, dans certains secteurs, rend de plus en plus difficile toute perspective de développement. Toutefois, selon nous, les solutions proposées dans ce texte ne répondent pas vraiment à la question de l'enclavement.

Dans son article 1, la proposition de loi donne un cadre, en fixant soit à 50 kilomètres la distance maximale d'accès à une unité urbaine, soit à une heure d'automobile l'accès à une ligne à grande vitesse. Je ne crois pas que ces critères répondent à l'enjeu du désenclavement des territoires. S'agissant du transport aérien, nous approuvons l'article 4 sur la qualité du service que doivent apporter les compagnies et l'exigence de résultat dont nous devons faire preuve. Enfin, je regrette que l'on traite du désenclavement sans évoquer plus largement le ferroviaire, qui peut pourtant apporter des réponses, tant à l'enjeu des mobilités qu'à celui de la transition écologique. Le désenclavement des territoires passe aussi par la lutte contre la fracture numérique. Au fond, en effaçant la notion de distance, le numérique a ouvert une nouvelle voie de désenclavement ; il a ouvert le champ des possibles pour les territoires ruraux. trop souvent, c'est l'inverse qui s'est produit. Dans les secteurs à faible densité de population, on s'est contenté de courir sans cesse derrière les avancées technologiques avec cinq ou dix ans de retard. Prenons le seul exemple de la couverture 4 G par l'opérateur Orange : on relève une couverture à 99 % pour les villes, contre seulement 39 % pour les zones rurales. Le numérique s'est donc installé en vecteur supplémentaire de l'enclavement des territoires. Nous le savons, la révolution numérique se poursuit. Elle nous ouvrira de nouveaux champs de développement, qui seront facteurs de désenclavement, à condition que nous sachions réussir ces nouveaux rendez-vous par une politique volontariste d'aménagement du territoire. Cet objectif mériterait d'être inscrit dans un texte de loi.

le premier facteur d'isolement des populations, donc d'enclavement. Je me trouvais la semaine dernière dans un secteur de mon département, un bassin de vie regroupé autour d'un bourg-centre, ancien chef-lieu de canton,

chers collègues, enclavement physique et numérique, isolement dans l'accès aux services essentiels à la vie quotidienne, ce sont bien des réponses globales que nous devons apporter pour réussir le désenclavement des territoires. C'est pourquoi nous regrettons

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier nos collègues du groupe du RDSE, en particulier Jacques Mézard, à qui j'adresse d'ailleurs mes félicitations pour sa récente nomination au Conseil constitutionnel, de nous permettre d'aborder aujourd'hui la question du désenclavement des territoires. En effet, la sénatrice des Hautes-Alpes que je suis peut témoigner des contraintes liées à l'absence de desserte routière, ferroviaire et aérienne dimensionnée dans un territoire rural et de montagne.

C'est donc au minimum douze heures de voyage par semaine. Cet exemple est d'autant plus significatif que le temps de trajet n'a cessé de s'allonger au fil des années en raison du nombre croissant de véhicules sur les routes, conséquence de l'augmentation des déplacements professionnels et personnels, sans que des solutions collectives adaptées soient proposées, voire sans qu'elles soient possibles, dans tous les départements. C'est aussi pour cette raison que la limitation de vitesse à 80 kilomètres par heure a été très mal vécue dans les territoires ruraux, où les habitants ont ressenti cette décision, venue d'en haut, comme une double peine, car, bien souvent, seule la voiture individuelle permet d'accéder à son travail, à la boulangerie ou à une unité de soins. Si la République française est une et indivisible, la France est diverse et plurielle. Ce texte nous offre donc la possibilité de rappeler qu'il n'existe pas une réalité territoriale, mais des réalités, et que les contextes économiques, géographiques ou sociologiques sont multiples. C'est pourquoi le droit à l'expérimentation doit être reconnu, plutôt que de remettre en cause ou casser ce qui fonctionne. La différenciation territoriale devrait enfin être une réalité pour les collectivités. En effet, faire confiance aux territoires, notamment aux présidents d'exécutifs départementaux, me paraît être une excellente chose, car nous en avons tous fait l'expérience : plus le centre de décision est éloigné, moins les décisions sont adaptées et comprises par nos concitoyens. Aussi, n'aurait-il pas été plus logique de laisser la limitation de vitesse à 90 kilomètres par heure et donner la liberté aux départements de fixer une vitesse maximale inférieure à celle qui est prévue par le code de la route, lorsque les circonstances En matière de sécurité routière, si la vitesse est un facteur aggravant en termes de risques, seules les modifications des comportements des automobilistes sur le long terme pourront agir de façon importante sur le nombre d'accidents mortels.

Dans ce domaine, un certain nombre de propositions ont été formulées par le Sénat et je me réjouis que les articles 5 et 6 les reprennent en partie, même si, une nouvelle fois, on peut regretter que les nombreuses mises en garde des sénateurs n'aient pas été entendues plus tôt par le Gouvernement et que ce texte ne vienne que rétablir ce qui existait auparavant. S'agissant de l'article 1 et de l'objectif de désenclavement à l'horizon 2025, il faudra se situer à moins de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile d'une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois. Si l'on peut se réjouir des précisions apportées aux critères de désenclavement, on peut craindre que la rédaction actuelle ne couvre que partiellement le territoire national. Je regrette pour ma part que, pour rompre l'isolement d'une ville ou d'un territoire, on se limite à l'aspect routier, car les objectifs ferroviaires ou aériens sont encore moins ambitieux. En outre, le désenclavement, ce sont aussi des services, je pense par exemple aux services de santé, en particulier aux maternités. Dans les Hautes-Alpes, une femme enceinte demeurant à Aiguilles, dans la vallée du Queyras, devra effectuer un trajet de plus d'une heure et dix minutes, dans le meilleur des cas, pour venir accoucher à la maternité de Briançon. Si l'objectif de désenclavement des territoires est louable et qu'il est l'une des principales batailles des sénateurs qui représentent la diversité du pays, il ne peut être atteint s'il ne s'accompagne pas d'une ferme volonté d'aménager le territoire ; deux notions pourtant essentielles pour retrouver l'unité de notre pays et renouer avec la solidarité nationale. Qu'en est-il de l'égal accès de chaque citoyen aux services publics, au savoir ou à la formation ? L'objectif fixé en matière de désenclavement est-il suffisamment ambitieux pour réduire la fracture territoriale et corriger les inégalités ?

: ceux qui sont privés de la capacité d'attirer des emplois, des services de santé ou des commerces, mais aussi les métropoles, qui connaissent parfois des situations d'asphyxie qui ne sont pas non plus très enviables. Et je ne parle pas de la saturation des

Je suis aussi convaincue- j'ai eu l'occasion de le dire en préambule, mais je veux le répéter -que la question des infrastructures est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut aussi être capable de proposer des services

François Bonhomme, sur l'article. L'article 1 souligne l'importance de prendre en compte l'objectif de désenclavement dans la programmation des investissements relatifs aux infrastructures de transport, ne serait-ce que pour répondre aux difficultés quotidiennes de nos concitoyens pour accéder à un emploi, à des services publics ou simplement à des biens de consommation essentiels. J'ajoute que cet enclavement est plus ou moins marqué selon les territoires. C'est une évidence ! Les rapports Les rapports du commissariat général à l'égalité des territoires nous rappellent régulièrement que les évolutions de long terme- désindustrialisation, vieillissement de la population, polarisation démographique ou métropolisation -sont des phénomènes majeurs, qui ont donné lieu à des évolutions territoriales très diverses et contrastées. Je ne veux pas opposer ici les métropoles dynamiques, captant les richesses et les opportunités, et les territoires périphériques délaissés, mais je crois que seul l'État

de désenclavement et de rapidité ... De ce point de vue, nous avons connu une véritable régression ! En quarante ans, des villes comme Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, Rennes ou Bordeaux se sont « rapprochées » de Paris. En revanche, En revanche, Toulouse et les territoires voisins sont les oubliés du plan TGV. La ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse pour relier Paris reste orpheline, alors même que, en quarante ans, les lignes à grande vitesse se sont développées dans les autres régions de France. dite POLT, a été négligée et que son entretien a largement fait défaut. Même si cet article peut paraître homéopathique, dans la mesure où il ne contient pas de principe actif, il a au moins le mérite de rappeler la nécessité pour l'État, même devenu impotent, d'investir de nouveau dans les infrastructures de transport et de prendre ainsi la mesure de la crise de l'aménagement du territoire que nous connaissons.

Déjà en 2014, dans son rapport sur l'hyper-ruralité, notre collègue Alain Bertrand posait parfaitement le diagnostic. Et le contexte dans lequel se trouve notre pays démontre que cet objectif a aujourd'hui toute sa pertinence. Nous connaissons la réalité des territoires les plus enclavés. Nous avons tous en tête des exemples d'usines qui ferment, de voies ferrées désaffectées, de routes dégradées, de services publics en recul. Je pense à la fermeture en 2008 de l'usine Molex dans dans le département de Françoise Laborde, qui a aussi touché une centaine de salariés du Tarn-et-Garonne, département de notre collègue Yvon Collin. Je pense aux menaces de fermeture de la gare de La Brillanne, dans le département de notre collègue Jean-Yves Roux, alors même que le trafic augmente. Je pense à ces villes moyennes, à ces centres-bourgs dévitalisés et à ces communes rurales, où le quotidien devient plus pesant. Nous connaissons bien sûr les efforts du Gouvernement, en particulier les vôtres, madame la ministre, mais il nous semble plus que jamais nécessaire d'accélérer le désenclavement des territoires grâce à un objectif national, afin de préserver nos infrastructures de transport et de les étendre. La voiture reste très souvent, au quotidien, le seul moyen de déplacement. C'est pourquoi nous proposons de rendre chaque partie du territoire métropolitain accessible à une autoroute,

à 2026. Cet objectif n'a rien d'irréaliste. Nous prenons d'ailleurs en compte la nécessité d'une cohérence de cet objectif avec la programmation régionale de l'aménagement du territoire, puisque les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les SRADDET, ne prendront en compte l'objectif qu'à compter de leur prochaine révision. Nos concitoyens attendent désormais du concret

du territoire, la lecture de l'article 1 a quelque peu douché mon enthousiasme ... En effet, cet article propose tout simplement de sortir la règle à calcul, afin de déterminer si, en tout point du territoire continental, une autoroute se trouve à moins de

au mieux, de s'arracher les cheveux, au pire, de baisser les bras ... Les élus locaux attendent plutôt du concret, en particulier de la part de leurs sénateurs.

Nous avons eu l'occasion de lui demander des précisions quant au calendrier de réalisation de cette infrastructure routière, qui est absolument indispensable. Il ne nous a pas répondu très clairement ... Nous enchaînons les contrats de plan, et ce chantier a

Ensuite, il restera un petit morceau de route qui est pratiquement en ligne droite. Il faut vraiment en finir. Nous en rediscuterons dans le cadre de la loi

: La parole est à M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à compléter l'objectif national de désenclavement créé par la proposition de loi, en sécurisant le lien de proximité entre les citoyens des territoires concernés et l'autorité préfectorale. Cet objectif permettra d'adapter les infrastructures de transport pour permettre à nos concitoyens d'atteindre une préfecture ou une sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. Les mouvements sociaux qui ont récemment traversé le pays nous ont montré dans l'imaginaire collectif, ce sont avant tout le maire et le représentant de l'État qui sont les premières institutions de dialogue pour l'ensemble de nos concitoyens. Or le lien et le contact direct avec l'administration préfectorale ont été sensiblement fragilisés depuis plusieurs années, années, avec les fermetures programmées de sous-préfectures, mais aussi avec la numérisation progressive de certains services de guichet- cartes grises, permis de conduire ... Comme l'a récemment souligné le Défenseur des droits- nous aurons tout à l'heure un débat sur la fracture numérique -, ces phénomènes posent problème pour les catégories d'habitants les plus fragiles, en particulier dans les territoires. Pour concilier la nécessaire modernisation de l'administration préfectorale avec l'impératif de proximité qui constitue son ADN, nous

de la réalité des territoires. Depuis la loi NOTRe de 2015, ce sont les régions qui gèrent l'essentiel des compétences en matière de transports et élaborent la planification des infrastructures. La loi d'orientation des mobilités, que nous examinerons prochainement, confère, quant à elle, une forte prégnance au couple intercommunalités-région. Toutefois, si les régions possèdent la robustesse financière et administrative nécessaire, leur nombre réduit a eu pour effet d'éloigner sensiblement les centres de décision des évolutions locales. Pour cette raison, il nous paraît pertinent d'associer à cette procédure le département et le préfet, qui restent des références en matière de proximité pour un grand nombre de nos concitoyens. La solution que nous proposons est juridiquement viable, puisque la région reste décisionnaire en matière de planification, mais pourra désormais bénéficier de l'expertise, de l'avis et des informations de cet échelon intermédiaire indispensable qu'est le département.

Quel est l'avis du Gouvernement ? La question du rôle respectif des intercommunalités, des départements et des régions dans la programmation des infrastructures de transports et le développement de services de mobilité est

témoigner à rebours de ce que je viens d'entendre. Tout d'abord, cet amendement est d'ores et déjà satisfait par l'article 10 de la loi NOTRe. Le département que j'ai eu l'honneur de présider a toujours pu trouver, dans l'espace régional, les instances de concertation nécessaires et suffisantes. Quant à ce transfert, je crois qu'il est illusoire de penser que nous allons défaire ce qui a été fait. Il nous revient,

puisque l'ensemble des personnels a gardé une résidence administrative au chef-lieu de département. Ce sont donc les mêmes fonctionnaires territoriaux qui assurent le service aujourd'hui. Tel est le témoignage que je voulais apporter pour expliquer mon abstention sur cet amendement.

Le scrutin est ouvert.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, voilà un mois, nous débattions des mobilités du futur et, à cette occasion, j'avais souligné les enjeux attachés, selon moi, au développement de l'hydrogène. C'est donc dans le prolongement de ce débat, mais aussi au vu de la question fondamentale de la transition énergétique pour notre pays, que le groupe du RDSE a choisi de mettre ce thème à l'ordre du jour du Sénat. Les opportunités qu'offre le développement de l'énergie hydrogène sont aujourd'hui documentées. Au regard de l'urgence écologique, elles doivent nous conduire à accélérer nos réflexions et nos décisions, afin de garantir le développement d'une filière d'excellence en la matière et d'accompagner le déploiement de cette énergie nouvelle, qui présente de multiples applications. L'hydrogène permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Convertible en énergie une pile à combustible, l'hydrogène peut en effet être utilisé dans les mobilités urbaines- voitures particulières, bus, trains -, le bâtiment ou encore l'habitat- production d'électricité et de chaleur. Il permet de développer la mobilité électrique dans l'ensemble du secteur du transport, un secteur utilisateur de 30 % de l'énergie consommée dans notre pays. L'hydrogène peut être facilement stocké et injecté, en étant par exemple associé au méthane, dans les réseaux de gaz naturel. Enfin, il représente un enjeu de compétitivité pour nos entreprises, à l'origine de nombreuses innovations. Oui, les initiatives existent déjà, et il faut les encourager J'en veux pour preuve l'action conduite dans mon département, le Pas-de-Calais, par le Syndicat mixte des transports Artois-Gohelle. Ce syndicat, qui couvre le territoire de trois agglomérations, représentant un demi-million d'habitants, lancera très prochainement sa nouvelle ligne de bus Les élus de ce territoire marqué par l'exploitation minière et une forte industrialisation ont fait le choix d'encourager le développement pour le réseau de transport en commun d'un mix énergétique. Ainsi, le réseau associera, à côté de bus circulant encore gasoil, des bus électriques et hybrides. Surtout, le syndicat lancera très prochainement une ligne assurée par des bus à hydrogène, la première de France, même si je sais qu'une réflexion similaire est en cours à Pau. Ces bus vont parcourir 420 000 kilomètres par an avec zéro CO2 rejeté, alors qu'un bus diesel Les élus ont également fait le choix de produire et de stocker l'hydrogène sur place en installant un électrolyseur, économisant ainsi le CO2 produit pour l'acheminement de l'hydrogène. La station rejettera, quant à elle, 374 tonnes d'oxygène, soit l'équivalent de 56 hectares de forêt. Les travaux de construction du dépôt se terminent, pour une ouverture dans les semaines à venir et une mise en circulation des bus cet été. Cet exemple illustre bien, madame la secrétaire d'État, le dynamisme de nos territoires. Il doit nous inspirer et pousser des initiatives similaires dans d'autres secteurs du transport comme l'aérien, le ferroviaire, le maritime ou le fluvial. Les technologies sont prêtes. Toutefois, nous le savons, le coût reste pour l'instant un facteur bloquant, et c'est là l'un des premiers défis auxquels nous sommes confrontés. Les coûts de fabrication peuvent pourtant être diminués en imaginant des mesures incitatives et en industrialisant la chaîne de production pour rentabiliser les investissements. saisirions ainsi l'occasion de développer une nouvelle filière industrielle créatrice d'emplois dans un contexte où notre tissu industriel est menacé, à l'image de notre filière sidérurgique, aujourd'hui en grande difficulté. Prenons aussi l'exemple du vélo à hydrogène, dont Mme Borne a parlé ici, voilà quelques semaines. Il s'agit d'une innovation de la société Pragma Industries, une première mondiale qui permet une autonomie de plus de 100 kilomètres, pour un temps de recharge d'une à deux minutes, quand l'électrique nécessite plusieurs heures.

Sur ce plan, le projet de loi d'orientation des mobilités aurait pu être plus volontariste, en intégrant par exemple des mesures incitatives pour accompagner le verdissement des flottes d'entreprises, de taxis ou de VTC, ou encore en étendant le forfait mobilité aux propriétaires des véhicules à très faibles émissions de CO2. Je veux néanmoins rendre hommage, ici, au ministre Nicolas Hulot, à l'initiative, en 2018, de notre premier plan hydrogène, lequel doit permettre, dès aujourd'hui, la mobilisation de 100 millions d'euros, dont une partie profitera à nos territoires les appels à projets de l'Ademe, à condition que les démarches administratives soient connues et simplifiées. L'un des trois axes de ce plan mérite plus particulièrement que l'on s'y arrête. Il s'agit de l'enjeu d'une production décarbonée de l'hydrogène. En l'effet, l'hydrogène porte l'ambition d'une énergie future totalement propre, mais à la condition qu'il soit produit lui-même, des énergies renouvelables. Les facilités qu'il offre en matière de stockage doivent notamment permettre une complémentarité avec le solaire et l'éolien, le stockage de l'énergie produite par ces moyens étant aujourd'hui complexe. Coupler des unités de production et de stockage d'hydrogène à des sites solaires ou éoliens représente un axe de développement et de réflexion dans notre recherche d'une énergie propre et renouvelable, seulement pour les transports, mais aussi pour le monde économique, qui a besoin d'énergie supplémentaire. Avec l'hydrogène, nul besoin de mettre en place des lignes aériennes supplémentaires qui défigurent le paysage. Là encore, les territoires nous montrent l'exemple. Nous connaissons tous le Grid, qui injecte de l'hydrogène dans le réseau de gaz de la communauté urbaine de Dunkerque, ou, à Paris, les taxis Hype. Hype. Plus simplement, un village de l'Aisne, Tupigny, a installé des éoliennes couplées à un électrolyseur qui produit de l'hydrogène, lequel est utilisé pour alimenter deux véhicules mis à la disposition des habitants pour réaliser leurs démarches administratives à la préfecture ou à la sous-préfecture. Toutefois, rien de structurant ne pourra se faire sans un engagement fort de l'État. D'ores et déjà, les acteurs de la filière mettent en garde sur la sécurisation des financements. Le premier appel à projets lancé par l'Ademe montre un nombre considérable de sollicitations, et toutes ne pourront pas être financées. Il est indispensable que l'État puisse dès aujourd'hui inscrire dans la durée ses financements et les majorer autant que nécessaire, car rien ne serait pire que de décourager les initiatives. l'AFHYPAC, appelle de son côté à la mobilisation de mécanismes de garantie des risques, notamment en cas de sous-utilisation des équipements, à l'image du dispositif France Transition, préconisé par le rapport Canfin-Zaouati. Oui, mes chers collègues, nous devons travailler pour forger un outil au service du renforcement des investissements, de la réorientation des flux privés, où l'argent public serait utilisé pour le partage du risque. La filière se trouve en effet confrontée à un déficit d'investissement et, si elle souligne l'existence de nombreux outils financiers, ils ne permettent pas, selon elle, de passer à l'échelle supérieure, c'est-à-dire à une véritable phase de déploiement. Il nous faut inventer des mécanismes de financement innovants, associant fonds publics et fonds privés, à l'instar de ce qui peut exister aux États-Unis ou au Japon, en couplant garanties, prêts bonifiés et fonds propres. Mes chers collègues, ce sujet est passionnant ; l'ambition est réelle ; l'enjeu en matière de développement durable est déterminant, d'autant que les technologies existent. Notre pays ne doit pas rater ce rendez-vous. Le recul récent annoncé par le Président de la République en matière d'objectifs de réduction de nos émissions de CO2 ne nous rassure pas, c'est peu de le dire. Le retard considérable que nous avons pu prendre sur des programmes innovants, comme les trains à hydrogène, est préoccupant.

de 2022-2024. Toutes les conditions sont réunies pour que nous avancions de façon unie sur le plan écologique et industriel, sans oublier les créations d'emplois qui pourraient en résulter. Ce dont nous avons besoin de toute urgence aujourd'hui, c'est d'une volonté politique forte pour accompagner ce tournant technologique que notre pays n'a pas le droit de manquer. À cet égard, madame la secrétaire d'État, nous en appelons à un engagement fort du Gouvernement. La parole

évoquer l'hydrogène aujourd'hui, c'est parler industrie, logistique, accessibilité, transport des personnes, énergie ou bien encore économie circulaire. Toutes ces activités recèlent des enjeux bien souvent imbriqués, qui font de l'hydrogène non seulement une solution crédible, mais surtout l'imposent comme un outil polyvalent, aussi bien face à un besoin ciblé que pour anticiper de nouvelles activités. Nos territoires, qui ont pleinement pris conscience des atouts de l'hydrogène, développent des projets innovants leur permettant de répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés : transition énergétique, qualité de l'air, aménagement du territoire et développement durable. Vous me permettrez donc d'articuler mon intervention à l'aune de l'expérience engagée- cela a été rappelé par Jean-Pierre Corbisez -sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, véritable terre d'hydrogène.

La communauté urbaine de Dunkerque est bel et bien dans le concret, en ayant choisi de pouvoir stocker l'électricité renouvelable sous forme d'hydrogène solide. En effet, le stockage de l'énergie issue des renouvelables est devenu une réalité. Le surplus de production d'électricité est désormais stocké sous forme d'hydrogène, une façon de résoudre les problèmes d'intermittence qui suscitent de plus en plus d'intérêt. C'est dans cette perspective qu'a été inaugurée, à l'été dernier, à Cappelle-la-Grande, située à quelques kilomètres de Dunkerque, une installation de dans un nouveau quartier de la ville. Le principe du est simple : il consiste à transformer l'électricité en hydrogène, qui peut, ensuite, être déstocké sur demande sous forme gazeuse, pour être injecté alors dans le réseau de gaz. En effet, l'hydrogène est probablement la meilleure façon de stocker l'énergie indéfiniment et sous forme solide. Cette technologie est une réponse à l'intermittence des énergies renouvelables, comme l'éolien ou le photovoltaïque, notamment en cas de surproduction en période de faible consommation, à l'origine de gaspillages énergétiques et d'une coûteuse surcharge du réseau électrique. La communauté urbaine de Dunkerque s'est lancée dans cette aventure en 2014, qui prend désormais la forme d'un démonstrateur installé dans la commune de Cappelle-la-Grande, collectant les surplus d'électricité produits par le parc éolien à proximité et par les panneaux photovoltaïques de la communauté de communes. Ce surplus d'électricité, transformé en hydrogène, est utilisé dans le réseau de gaz naturel, alimentant ainsi 200 logements. On voit là l'intérêt de l'hydrogène issu des renouvelables, qui est de décarboner le gaz naturel et de permettre de réduire les émissions de CO2, d'améliorer la qualité de l'air et d'augmenter nettement les rendements des chaudières à condensation de 7 % à 10 %. Ce démonstrateur fonctionnera pendant deux ans, en conditions réelles, sans surcoût pour les utilisateurs. La part d'hydrogène dans le gaz naturel a d'ailleurs été augmentée progressivement. De 6 % en juin 2018, elle est passée à 20 % en janvier 2019, soit le seuil le plus élevé testé en Europe. Ces années vont permettre d'analyser la réaction du matériel, notamment les éventuels problèmes de corrosion des chaudières, le pouvoir calorifique du mélange gaz naturel hydrogène, mais aussi l'acceptabilité du procédé par le consommateur et sa viabilité économique. Cette expérimentation est bien l'illustration que la transition énergétique s'opère sur nos territoires, mais aussi dans le cadre de cette stratégie nationale en plein essor. Ce projet, qui est le beau symbole de mutations, doit en permettre d'autres, s'inscrivant pleinement dans le cadre du plan hydrogène présenté en juin 2018- cela a aussi été souligné par Jean-Pierre Corbisez. Comme le Comme le rappelle régulièrement le maire de Dunkerque, la transition énergétique se fait dans les territoires. On n'a pas envie de la subir, et ce projet un beau symbole des mutations parlant d'hydrogène, alors que nous allons entamer, le 19 mars prochain, la discussion du projet de loi d'orientation des mobilités et que la ministre Élisabeth Borne était parmi nous il y a encore quelques instants, vous me permettrez d'évoquer plus particulièrement les enjeux de l'hydrogène en matière de mobilité. Élisabeth Borne le rappelait le 1 juin 2018, l'hydrogène apportera sans aucun doute une part importante des réponses pour décarboner et dépolluer nos solutions de mobilité. Nous le savons, l'hydrogène embarqué apporte en effet pour l'électromobilité des solutions nouvelles concernant en priorité les véhicules à usage professionnel, qu'ils soient terrestres, maritimes, fluviaux ou ferroviaires. La mobilité hydrogène fait déjà l'objet de développement concret avec les taxis et les bus. L'enjeu pour la mobilité de demain, sur laquelle nous reviendrons dans nos débats, est de favoriser dès aujourd'hui le passage à l'échelle, comme l'a rappelé l'intervenant précédent. En matière ferroviaire, nous avons là de véritables objectifs qui ont fait l'objet d'un rapport déposé par un député sur le verdissement du ferroviaire. Nous le voyons bien, l'hydrogène est, sans conteste, une ressource avec laquelle il faut compter dans le cadre d'une transition transition écologique réussie. Là aussi, les débats que nous aurons lors de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités nous permettront de mesurer que le mix énergétique, s'agissant de mobilité, est essentiel pour proposer des solutions décarbonées.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ce débat, demandé par le groupe du RDSE, que nous remercions, s'inscrit complètement dans l'actualité, tant il y a une urgence à trouver des alternatives aux énergies carbonées. Certes, il ne s'agit pas de penser naïvement que l'hydrogène sera le carburant de l'économie de demain, l'élément miracle qui nous détachera de notre monde fossile et fissile ! Toutefois, ses potentialités sont indéniables. De quoi parlons-nous ? L'hydrogène est un gaz connu, déjà utilisé par l'industrie pour fabriquer des engrais, raffiner des carburants et destiné à de multiples usages plus ponctuels, comme le lancement des fusées. En termes énergétiques, l'hydrogène constitue un vecteur stable, qui peut être stocké, à la différence de l'électricité, même s'il faut manipuler de gros volumes- quatre fois ceux du gaz naturel. Ainsi, et c'est tout l'enjeu, associé aux piles à combustible, l'hydrogène pourrait être utilisé beaucoup plus largement à l'avenir comme vecteur d'énergie pour les transports et la production d'électricité. L'électricité ainsi produite peut donc faire tourner un moteur, par exemple celui d'une voiture électrique, avec un bon rendement, sans bruit, avec émission de chaleur, mais sans dégager de gaz polluant. C'est pourquoi beaucoup voient aujourd'hui en cette évolution une révolution aussi importante que celle qui fut provoquée par l'utilisation du charbon au début de notre ère industrielle. Comme le soulignait Nicolas Hulot dans sa présentation du plan hydrogène : « C'est aujourd'hui la seule technologie qui permette de stocker massivement et sur de longues périodes l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables intermittentes. C'est donc un élément clé de la stabilité du mix électrique de demain. Certes ! Mais cette utilisation énergétique de l'hydrogène ouvre de nouvelles questions et pose quelques problèmes. Tout d'abord, la production occasionne des émissions de CO2 ou, dans le cas de l'électrolyse, nécessite de grandes quantités d'électricité. Ensuite, s'agissant de son transport et de son stockage, il faut faire appel à des dispositifs spécifiques, à haute pression ou à très basse température, qui sont chers, lourds et encombrants. Enfin, en ce qui concerne son utilisation, on a besoin de piles à combustible qui coûtent très cher, s'usent rapidement et requièrent une grande quantité de métaux précieux. Cela étant, toutes les pistes alternatives aux énergies fossiles doivent être sérieusement explorées. Comment faire pour que cela fonctionne ? Alors que le Gouvernement a fait le choix d'un État régulateur plutôt que d'un État interventionniste, ce débat sur l'hydrogène comme énergie d'avenir nous rappelle que sans intervention publique forte, il n'y aura pas de transition énergétique à la hauteur des enjeux climatiques d'aujourd'hui. de l'énergie, l'Ademe : « Le déploiement d'une filière hydrogène nécessite des investissements relativement lourds, tant pour la production, la distribution que le stockage de l'hydrogène. Ceux-ci supposent un engagement d'acteurs industriels et une maîtrise du risque économique par le soutien des pouvoirs publics En effet, tout comme le déploiement des réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphonie, les nouveaux systèmes énergétiques basés sur l'hydrogène auront un coût de démarrage élevé, et ils présentent une incertitude quant à l'évolution de la demande. Il est donc peu probable que les entreprises privées investissent seules dans l'infrastructure nécessaire pour élargir l'utilisation de l'hydrogène à l'échelle nationale. De plus, les consommateurs ne pourront acheter une voiture à hydrogène que s'il y a une infrastructure suffisamment dense de stations de distribution du carburant. En effet, l'ouverture de stations d'hydrogène en dehors des grandes villes sera un facteur déterminant pour la diffusion des carburants alternatifs, mais les acteurs privés se concentreront naturellement sur les zones rentables. C'est pourquoi nous pensons que seul l'État peut jouer un rôle décisif pour la mise en place des infrastructures, ce qui permettrait de sortir du « cercle vicieux » qui empêche le démarrage de la filière. Dans le cas d'une innovation radicale comme l'hydrogène, l'intervention publique est indispensable, d'une part, pour soutenir la technologie pendant la phase qui précède l'entrée dans le marché sur les questions de recherche, de développement et de démonstration, de manière à la rendre compétitive face aux technologies conventionnelles, d'autre part, pour aider l'innovation à entrer sur le marché, notamment en soutenant les investissements dans l'infrastructure. Or cette intervention est actuellement limitée par la situation budgétaire des gouvernements et la conception de l'État, plus perçu en régulateur de l'activité économique qu'en investisseur. Comme le souligne l'Ademe : « Le recours au vecteur hydrogène apportera des solutions, de la flexibilité, des services pour la mise en oeuvre de la transition énergétique, mais il ne peut conduire à limiter les efforts à engager, notamment en termes de maîtrise des besoins et d'efficacité énergétique. Une forte diminution de la consommation de combustibles fossiles est vitale, et elle passera, certes, par le développement des autres ressources. Il ne faut cependant pas se voiler la face, la dépendance à l'égard du pétrole ne peut être durablement réduite qu'en limitant la place de la voiture individuelle au profit des transports en commun. Il faut maintenant parler de leur gratuité. Il faut aussi penser à l'urbanisme différemment, par exemple, en rapprochant le lieu de travail du domicile et supprimer ainsi les trajets quotidiens énergivores. Il faut enfin que l'État réinvestisse dans le fret ferroviaire, qui, malgré tous les grands discours, ne cesse de reculer. Bref, il faut un diagnostic, mais aussi une vision d'avenir et une intervention globale de l'État ; aujourd'hui, malheureusement, nous en sommes bien loin ! La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je remercie, tout d'abord, le groupe du RDSE de la tenue de ce débat sur un sujet très intéressant et important au regard des enjeux de l'actualité. l'heure où le glacier Thwaites, en fusion à cause du réchauffement climatique, menace de rendre plus que réel le risque de submersion des côtes du monde entier, phénomène proprement catastrophique et inédit, nous devons absolument et rapidement mettre en place des solutions pour réduire les gaz à effet de serre, les deux principaux étant le méthane et le dioxyde de carbone. Nous sommes en effet à la croisée des chemins et devons faire des choix responsables pour l'avenir afin d'éviter l'irréversibilité du changement climatique. Il y a, en cela, urgence absolue En la matière, l'hydrogène est un fabuleux espoir. C'est un gaz incolore et inodore, très léger, combustible, donc, capable de libérer par combustion de la chaleur et de l'énergie. Lors de cette réaction chimique, il ne produit que de l'eau sous forme de gaz, c'est-à-dire de la vapeur d'eau. Il présente un potentiel extraordinaire pour répondre à nos enjeux de transition énergétique, mais il n'existe pas dans la nature. L'enjeu, aujourd'hui, serait de le produire de manière décarbonée, c'est-à-dire sans sans la technique jusqu'à présent utilisée de vaporeformage du méthane, laquelle génère de l'hydrogène que l'on pourrait qualifier de « gris ». Au contraire, on peut produire de l'hydrogène par électrolyse, en faisant passer du courant électrique dans de l'eau. Il se produit alors des réactions chimiques au niveau des électrodes et il se forme, à la cathode, du dihydrogène. Ce procédé coûteux, au rendement très moyen, n'a été jusqu'à présent que peu utilisé. Si on développe les énergies renouvelables, on peut avoir la solution. La production d'électricité des éoliennes et des panneaux photovoltaïques est variable. En revanche, elle peut atteindre des pics, notamment en été, à des heures où la demande est moins importante. Cette électricité produite pourrait alors alimenter les électrolyseurs et produire un hydrogène « vert Actuellement, la recherche se développe et les résultats s'annoncent d'ores et déjà prometteurs. Le CEA-Liten à Grenoble travaille sur la technologie SOEC, électrolyse à haute température et à haut rendement, en vue de son industrialisation dans un avenir très proche- on parle de cinq ans.

Il suffit d'équiper un véhicule d'une pile à combustible. Dans cette pile, l'hydrogène fournit de l'électricité en ne produisant, comme je l'ai dit, que de la vapeur d'eau. J'ai pu voir fonctionner un bus utilisant cette technologie à Cologne, en Allemagne. À terme, c'est tout le réseau de cette métropole qui roulera à l'hydrogène. Le réservoir se remplit rapidement- c'est un réservoir à hydrogène. Sa capacité est équivalente à celle d'un véhicule diesel, et il possède donc en cela une grande autonomie. Les avantages ne s'arrêtent pas là, le moteur étant plus puissant qu'un moteur classique électrique. Cette technologie pourrait être l'avenir de nos poids lourds, mais aussi des trains fonctionnant sur des petites lignes non électrifiées. Le scénario exposé par le projet du « verdissement du parc ferroviaire » fixe à 2035 le remplacement de trains régionaux roulant au gazole par des trains roulant à l'hydrogène. Cette perspective de 20 % de déplacements propres sera, je l'espère, tenue. Pour ce faire, les énergies renouvelables doivent se développer. Selon RTE, notre stade de développement est actuellement insuffisant. Du volontarisme est absolument nécessaire, car nous avons du retard C'est de la création d'un réseau énergétique supplémentaire qu'il est question. Il faudra consentir des efforts d'investissement et accepter d'entretenir des infrastructures qui n'existent pas aujourd'hui. Le plan Hydrogène est ambitieux, très engageant, mais il doit passer à une phase de réalisation plus offensive. Il faudra que tout le territoire national soit concerné pour que cela vaille la peine. Peut-on en rester à de simples appels à projets et laisser au bon vouloir des uns et des autres le loisir de faire ou pas ? En cela, je crois que l'État devrait reprendre son rôle de stratège. La parole

vers des modes de production durables, sobres, mais aussi de plus en plus décarbonés. Année après année, nous disposons de rapports à leur tour sans cesse plus réalistes, qui nous exhortent à accélérer des investissements directs en faveur de cet objectif : rapport du GIEC de septembre 2018, en tête. La stratégie climat de la Commission européenne, communiquée en novembre dernier, semble, elle aussi, vouloir passer à la vitesse supérieure, puisqu'elle pose le principe d'une neutralité carbone de l'Europe en 2050. Ici, en France, une pétition a réuni près de deux millions d'habitants, pour proposer une plus grande visibilité de la stratégie nationale et européenne. Dans ce contexte, où il ne s'agit plus de tergiverser, l'hydrogène apparaît comme une possibilité intéressante en vue d'accompagner cette trajectoire, en particulier, là où, de l'avis même du commissaire européen au climat, notre pays est en retard sur ses objectifs, l'augmentation de la part d'énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Il s'agit évidemment non de fournir une recette miracle, mais de vivre pleinement une opportunité industrielle, sociétale et environnementale majeure. À ce titre, nous devons garder en mémoire les débats qui se sont tenus au moment de l'exploitation possible des gaz de schiste, exploitation abandonnée en Grande-Bretagne, abandonnée en Pologne, jugée écologiquement et économiquement Nous disposons aujourd'hui d'une connaissance précise des multiples possibilités de l'hydrogène, de son traitement et de l'exploitation dans des conditions décarbonées. Il s'agit, tout d'abord, de produire des technologies alternatives vertes pour des industries très consommatrices d'hydrogène. Parmi les applications les plus visibles, on trouve l'équipement de modes de transports lourds et la mise en circulation de flottes de véhicules à hydrogène, avec des stations de recharge correspondantes. Le 1 juin dernier, le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, a annoncé la mise en oeuvre d'un plan hydrogène doté, en principe, de 100 millions d'euros par an jusqu'en 2023- en réalité, de 100 millions d'euros en 2019 -, avec une évaluation du niveau de déploiement des industries. Le ministre a ainsi affirmé, que dans la perspective de la transition énergétique, « l'hydrogène peut aussi devenir une solution majeure pour notre énergétique tout d'abord en rendant possible le stockage à grande échelle des énergies renouvelables, permettant ainsi de rendre crédible un monde où l'hydrogène vient se substituer, petit à petit, au fossile et au nucléaire pour combler les intermittences du solaire et de l'éolien Ce plan donne, par ailleurs, à la filière hydrogène deux missions principales : tout d'abord, stocker l'électricité produite par des filières renouvelables intermittentes sous forme d'hydrogène produit par électrolyse de l'eau, ensuite, distribué dans un réseau de gaz ou utilisé dans une pile à combustible pour produire de l'électricité, ensuite, ensuite, développer des « mobilités propres », en utilisant l'hydrogène dans une pile à combustible alimentant un moteur électrique. Ce plan, qui doit donner lieu à un accompagnement important de l'Ademe, est assorti d'une aide directe à l'acquisition d'électrolyseurs, d'aides à la mise en place de projets territoriaux pilotes en matière de mobilité, aide sous forme d'avances remboursables pour les stations de recharge et de l'aide à l'acquisition de véhicules professionnels ou de véhicules destinés au transport collectif. Enfin, ces aides pourraient être mobilisées dans des zones non interconnectées aux réseaux, associant plusieurs usages de l'hydrogène. Madame la secrétaire d'État, 2019 est, de fait, une année d'amorçage et de pari industriel, qui suscite de fortes attentes et espoirs chez les acteurs de la filière, mais aussi chez les collectivités locales. Ce plan, mes chers collègues, demande de la constance, du temps et une stratégie. Les industriels, comme les acteurs de la filière, ont en effet besoin, pour pleinement se déployer, d'assurances et de moyens à long terme. Je souhaite rappeler, madame la secrétaire d'État, que des territoires ont d'ores et déjà effectué ce pari industriel et énergétique. Outre les vingt-neuf projets « territoires hydrogène » sélectionnés et mis en oeuvre en 2016, d'autres EPCI se sont dotés de stratégies de diversification énergétique à grande échelle. Dans ce contexte, vous permettrez, madame la secrétaire d'État, que nous soyons attentifs à la forte visibilité de la mise en oeuvre des projets sélectionnés dès cette année. L'enjeu est bien d'engager des projets qui permettront, dès à présent, de faire baisser le coût de l'hydrogène et de lancer la fabrication et la commercialisation de piles à combustible par les industriels. Or cet enjeu demande, à n'en pas douter, une structuration plus importante de l'ensemble de la filière hydrogène. Au total, nous plaidons pour que la mise en oeuvre du plan hydrogène soit visible et accessible, et ce dans tous les territoires, urbains comme ruraux, avec des applications concrètes. en effet de la visibilité des projets que dépendra le contrat social et environnemental qui liera nos concitoyens, déjà éprouvés par une facture énergétique lourde pour les petits revenus, aux objectifs même de la transition énergétique. La parole

Une actualité marquée par la proclamation du président Macron, après la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, et son souhait affiché de faire de notre pays le leader mondial pour le climat. Une actualité affectée, j'y reviendrai, par diverses crises industrielles. Enfin, notre échange d'aujourd'hui nous permettra assurément de nourrir notre réflexion avant que nous n'examinions le projet de loi sur les mobilités. Tout cela impose aux parlementaires que nous sommes de chercher le nécessaire équilibre entre la réduction des émissions des gaz à effet serre et la vitalité économique, sans, en explorant toutes les pistes envisageables.

Il pourrait alors occuper une place de choix dans la transition énergétique. Rappelons que l'hydrogène est l'élément le plus simple et le plus léger que l'on trouve dans notre univers. Il ne se compose que d'un seul proton et d'un seul électron. L'hydrogène est aussi l'élément le plus abondant : 75 % en masse et plus de 90 % en nombre d'atomes. Cependant, la molécule d'hydrogène, H2, n'est plus jamais seule. Elle est toujours combinée à un autre élément comme l'eau, H20, ou le méthane, CH4. L'hydrogène, qui est aujourd'hui principalement utilisé par l'industrie, est malheureusement produit à 95 % à partir de combustibles fossiles. Dans le contexte de la transition énergétique, l'enjeu majeur est donc de décarboner la production de l'hydrogène. Je vous rappelle que le Gouvernement a doté la France de l'objectif ambitieux d'atteindre, en 2050, la neutralité carbone, entendue comme l'atteinte de l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions anthropiques- forêt, prairies, sols agricoles, zones humides ... -à l'échelle territoriale. Pour cela, il est nécessaire que le système énergétique évolue, afin que les énergies consommées sur le territoire français n'émettent plus de gaz à effet de serre. Dans son action, le Gouvernement s'appuie sur la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui décrit la feuille de route de la France pour conduire la politique d'atténuation du changement climatique. également sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, qui fixe les priorités d'actions des pouvoirs publics dans le domaine l'énergie. Cette programmation inscrit la France dans une trajectoire qui, je vous le rappelle, mes chers collègues, doit nous permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Dans les différentes programmations publiées par le ministère de la transition écologique, l'hydrogène décarboné fait partie des gaz renouvelables qui doivent, en 2050, fournir 180 térawatts au pays. Une grande ambition, donc, pour une énergie qui apparaît comme inépuisable. Il faut néanmoins que nous soyons vigilants. En effet, l'hydrogène ne peut être produit qu'à partir de deux procédés. à partir d'énergies non renouvelables, c'est-à-dire d'hydrocarbures et de charbon. Aujourd'hui, 95 % du dihydrogène produit découle de cette méthode.

Encore une fois, il convient de ne pas être hypocrite. Il est en effet nécessaire que l'hydrogène soit produit à partir d'une électricité qui soit elle-même décarbonée ou produite à partir d'énergies renouvelables- outre l'éolien et les photovoltaïques, déjà cités, n'oublions pas les barrages.

Ainsi, il apparaît clairement que l'hydrogène se présente comme une énergie d'avenir si nous parvenons à en assurer la production et le stockage, évidemment à partir d'énergies renouvelables. Alors que la première voiture grand public à hydrogène a été mise en service dès 2014, alors que l'Allemagne développe cette énergie renouvelable depuis le début des années 2010 et a investi pour cela près de 1,4 milliard d'euros, alors que la Chine a démarré un investissement de 8 milliards de dollars dès 2015, la France connaît, reconnaissons-le, un large retard en la matière. Nous envoyons déjà des fusées dans l'espace grâce à l'hydrogène. Je rappellerai d'ailleurs que les satellites qui ont amené en 1969 les hommes sur la lune fonctionnaient avec des piles à combustible.

Le principe est simple : l'énergie est utilisée pour produire du dihydrogène, H2, le plus souvent sous pression. Puis, ce dihydrogène peut, soit alimenter une pile à combustible, libérant de l'électricité, soit être brûlé directement, produisant une énergie calorifique. Les applications s'orientent sur deux axes. Le premier est de stocker de l'hydrogène pour le convertir en électricité. De nombreuses expérimentations sont en cours, comme en Guyane, où se construit la plus grande unité de stockage du monde fonctionnant sur ce principe.

développer plus rapidement ce système pour d'autres types de véhicules. Associé à un moteur électrique, il peut offrir des rendements plus élevés qu'une batterie Lithium-Ion, produisant nettement moins de pollution. Cela explique la frénésie de recherche dans cette technologie, notamment pour l'automobile et le transport ferroviaire. À ce sujet, un député du Médoc, M. Benoît Simian, avait préconisé, à l'occasion d'un rapport qu'il a remis à Mme Élisabeth Borne, la mise en place de trains roulant à l'hydrogène vers 2022.

Vous le savez, depuis la loi NOTRe, les régions françaises se sont pleinement saisies de cette question. Par exemple, la région Nouvelle Aquitaine s'associe, pour 3 millions d'euros, avec les régions Grand Est et Occitanie au projet de développement d'un TER hybride avec stockage d'énergie embarqué, porté par la SNCF.

Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisables. » À nous de saisir cette chance

je souhaite vous faire part de nos réflexions sur l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie d'avenir. La molécule d'hydrogène a de nombreuses qualités. Il a souvent été question de sa vertu écologique : son utilisation ne pollue pas.

cette molécule apparaît de plus en plus pertinente comme source d'électricité. Associée à une pile à combustible, elle remplit le rôle de batterie, ce dans tous les domaines, du transport jusqu'à l'habitation. divers projets sont en cours dans les secteurs du transport maritime et aérien, notamment grâce à une entreprise très importante, la société Safran. En matière ferroviaire, le premier train commercial à hydrogène, construit par un constructeur français, Alstom, circule déjà en Allemagne. Pourquoi ne circule-t-il pas encore en France ?

la production d'hydrogène avec de l'eau et du courant électrique : c'est une solution très intéressante pour lisser la production renouvelable d'électricité, qui a très souvent la faiblesse de l'inconstance. nous saluons l'initiative du village de La Nouvelle, situé sur l'île de la Réunion, qui expérimente déjà un tel mix énergétique. L'un des principaux freins au déploiement de cette technologie reste son coût très élevé. L'hydrogène ne connaîtra pas de développement rapide et ne donnera pas tous ses fruits sans investissements d'ampleur, et c'est tout à fait normal. D'une part, ce gaz est très volatil, très inflammable et explosif, ce qui est de nature à rendre complexes et chers sa production, son acheminement et sa distribution- mais l'industrie française a déjà réglé des problèmes la fabrication de la pile à combustible reste très onéreuse en raison du platine qu'elle exige. Il nous semble qu'une politique d'aménagement et d'infrastructures, en garantissant des conditions de sécurité maximales, pourrait favoriser l'utilisation de cette technologie. Ainsi, des économies substantielles pourraient être réalisées en utilisant l'hydrogène, afin d'éviter la coûteuse extension de lignes électriques pour alimenter des territoires ou des voies ferrées isolés : on le sait, de tels

Ce vecteur d'énergie aura certainement un grand rôle à jouer dans le mix énergétique de demain ; naturellement, cette transformation ne devra pas être accomplie au détriment de la sécurité. Il faudra donc prendre toutes les précautions

bienvenu. La question de l'hydrogène se pose à présent de manière préoccupante- je pense en particulier au remplacement de l'hydrogène gris utilisé par nos industries, peu coûteux, mais très polluant, par de l'hydrogène vert décarboné. En outre, l'hydrogène a pleinement son rôle à jouer dans la mobilité, dans la transition énergétique et écologique des transports. Nicolas Hulot l'an dernier, contient un volet « décarbonisation de l'hydrogène industriel », un volet « mobilité » et un volet « stockage ». Il vise donc bien à structurer la filière et à participer au mix énergétique. Une enveloppe de 100 millions d'euros a été annoncée et confirmée dans la Mais cet ensemble de mesures n'est pas à la hauteur des enjeux industriels et écologiques français et internationaux. En effet, sur le plan industriel, la production d'hydrogène vert en remplacement de l'hydrogène carboné très polluant est à présent possible et parfaitement définie d'un point de vue technologique, grâce notamment à la biomasse, mais surtout à l'électrolyse de l'eau. Ce peut tout aussi bien s'appliquer aux camions, aux bus, aux trains, aux voitures, etc. Le gros avantage de l'hydrogène est son pouvoir de stocker les énergies renouvelables éolienne, photovoltaïque et hydroélectrique, produites en discontinu, mais rarement aux moments de grosse consommation. L'enjeu est donc majeur au regard de la transition énergétique. Jusqu'alors, les seules solutions de stockage étaient les barrages hydrauliques et les stations La filière « » permettra un stockage massif, une activation flexible et une restitution polyvalente. Les énergéticiens tels qu'EDF, Engie ou Total s'y intéressent d'ailleurs aussi. Lors de sa visite en Savoie en janvier dernier, Mme Brune Poirson a pu constater les avancées technologiques de l'entreprise Atawey. D'autres start-up sont aussi dans les starting-blocks, si je puis m'exprimer ainsi. Des industriels sont prêts : je pense par exemple à l'entreprise H2V, qui a pour ambition de produire dans ses usines, à coût moindre que l'hydrogène gris, jusqu'à 200 000 tonnes d'hydrogène vert, de développer une véritable filière industrielle et de créer 12 000 emplois en France d'ici à 2025.

Les surcoûts inhérents à toute nouvelle technologie restent élevés. Aussi, le plan doit absolument créer les conditions d'investissements industriels susceptibles de permettre la baisse des coûts, par complémentarité entre l'action publique et les porteurs de projets privés. de régulation de l'énergie, la CRE, pour ce qui concerne l'hydrogène, dans le cadre de la PPE. Il semblerait que personne n'ait pris en main cette organisation de base pour que soient développés des prix encadrés et réglementés, indispensables pour les industriels.

il pourrait être judicieux de mettre en oeuvre un dispositif de garantie d'origine permettant de caractériser l'hydrogène renouvelable et son intérêt décarboné. Au surplus, il est nécessaire d'accompagner la transformation des métiers par la formation continue, afin d'orienter les emplois existants des filières industrielles et techniques vers la filière hydrogène. Une entreprise française a déjà développé des programmes de formation spécifiques, en collaboration avec les régions et les universités, pour préparer la nouvelle « génération hydrogène » et relever les défis actuels.

Ces dernières permettent une recharge des véhicules aussi rapide que de faire un plein en carburants classiques, à des coûts qui pourront être inférieurs. Leur déploiement permettra de résoudre la double équation du pouvoir d'achat et de la protection de notre environnement. Pour conclure en quelques mots, si l'hydrogène est bel et bien une énergie d'avenir, s'il a toute sa place dans le mix énergétique en permettant le stockage de l'électricité renouvelable et une mobilité décarbonée, il est indispensable d'accélérer les démarches législatives et réglementaires pour permettre à nos industriels français de monter en puissance en la matière. Cette filière d'excellence, prête à se développer, ne doit pas nous échapper au profit de nos concurrents européens et internationaux.

Face à l'urgence climatique, faut-il apporter des corrections à la marge ou nous donner une chance pour demain, en préparant cette mutation indispensable qu'est la décarbonation de notre économie ? Les pays qui se préparent doivent dès maintenant promouvoir une authentique filière hydrogène, grâce à un plan d'investissements massifs à court, moyen et long termes. Il s'agit bien de fabriquer de l'hydrogène décarboné à partir d'énergies douces. Rappelons tout de même que la mutation énergétique de l'hydrogène apporte ce qui manque cruellement aux énergies renouvelables : des capacités de stockage. La filière hydrogène peut permettre un développement inédit

: vous faites ce choix au moment où la Californie prévoit 100 stations hydrogène pour 2020 ; au moment où le Japon crée un consortium de ses fabricants automobiles pour un passage rapide à l'hydrogène, dès les années qui viennent, même si l'hydrogène

Certes, nous nous battons pour une usine européenne de batteries ; mais avouez que nous sommes loin du compte pour ce qui concerne l'emploi. Garder des choix technologiques ouverts, c'est préserver les possibles, c'est refuser de se refermer sur une seule stratégie, c'est écarter des choix totalisants. Le moteur atmosphérique peut encore être dépollué très sensiblement et consommer beaucoup moins. L'électrique prendra une part, mais elle sera limitée. Prenons garde : la Chine va présenter un véhicule électrique à 8 500 euros, grâce à de nombreuses subventions d'État.

Madame la secrétaire d'État, ne retardez pas la décarbonation de notre industrie. Cette filière est un élément fondamental, avec l'industrie du futur, pour réindustrialiser la France, pour réindustrialiser l'Europe.

je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisables. » À nous de saisir

Aujourd'hui, alors que nous nous demandons encore s'il est judicieux de développer les technologies autour du vecteur hydrogène, j'ai le sentiment que nous ne sommes plus capables d'audace scientifique ; que la capacité de rêver, propre à Jules Verne, s'est largement émoussée que l'enthousiasme suscité par la potentialité de découvertes disruptives s'est éteint. Pis, coincée entre les intérêts bien sentis que défendent les uns et les craintes peu propices au changement qu'éprouvent les autres, notre recherche semble au point mort, dans un champ pourtant désigné depuis des décennies comme l'avenir de notre production énergétique. Après un siècle et demi d'exploitation industrielle du pétrole, dont on nous dit que les réserves mondiales s'amenuisent, nous devons nous interroger en profondeur : quelle est la meilleure source énergétique pour alimenter notre industrie, pour fournir la chaleur aux bâtiments publics et aux habitations particulières, pour faire fonctionner nos avions, nos bateaux, nos trains et nos automobiles- toujours plus nombreuses -, lesquelles provoquent une pollution atmosphérique qui n'est plus soutenable dans un certain nombre de mégalopoles Partout dans le monde, à la fois pour des questions de ressources et pour des préoccupations environnementales, se profile une massification du véhicule électrique. Il nous faut réinventer notre production d'électricité : celle de demain ne ressemblera vraisemblablement pas à celle d'hier. Dans cette perspective, la filière nucléaire, si caractéristique de l'indépendance énergétique de notre pays, a toute sa place : elle ne doit évidemment pas être abandonnée. Au contraire, nous devons consolider notre savoir-faire, qui progresse notamment avec l'émergence de nouveaux procédés de traitement des déchets radioactifs, et envisager de nouvelles unités de production, aux dimensions peut-être plus modestes que les précédentes. Parallèlement, nous ne pouvons plus négliger, pour notre futur mix énergétique, ce pan entier que constitue l'hydrogène, élément à la fois si présent dans la nature et si difficile à isoler. La possibilité de le stocker et de le diffuser rapidement constitue des atouts indéniables. Bien sûr, je ne méconnais pas les reproches qui sont adressés à la production d'hydrogène par reformage du méthane ou par électrolyse de l'eau. On dénonce, essentiellement, son bilan carbone aujourd'hui extrêmement défavorable. de substitution se font jour : il s'agit par exemple d'associer en amont une méthanisation, qui est une réelle chance à saisir pour nos territoires et nos agriculteurs. Je crois surtout que le génie humain est capable de surmonter ce type de difficultés. Encore faut-il déployer des moyens en adéquation avec les ambitions ; encore faut-il définir une véritable stratégie de long terme, susceptible d'enclencher, par une sorte de ruissellement, une véritable dynamique et,, de donner les résultats attendus.

Avec 100 millions d'euros par an, pendant cinq ans, pour un chantier d'une telle ampleur, et comparativement à ce qui se profile dans d'autres pays, on ne peut raisonnablement pas imaginer que nous sommes engagés vers une véritable transition énergétique.

La défiance qui s'exprime actuellement envers les élus nous ordonne d'assumer nos missions, de donner un cap au lieu de porter des coups, de mettre à profit l'expertise qui nous entoure plutôt que de la jeter aux orties.

orienté exclusivement vers le véhicule électrique à batterie, alors que nombre d'avis expriment nettement la nécessité de diversifier notre approche des futures mobilités propres. Enfin, cessons de dire, à grands renforts médiatiques, que nous pouvons, seuls, bouleverser les choses et inventer un nouveau modèle énergétique. Dans trois mois se dérouleront des élections européennes. Je veux croire que les programmes prochainement dévoilés feront la part belle à un projet européen susceptible de rivaliser avec les grandes manoeuvres observées, en particulier, en Chine. Emmanuel Macron, a annoncé un Airbus de la batterie, avec une participation de 700 millions d'euros pour la France ; grand bien lui ferait de s'engager plus nettement encore sur la voie du développement de la filière hydrogène.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en prenant connaissance de l'intitulé de ce débat, « L'hydrogène, une énergie d'avenir »,

En définitive, l'hydrogène ne serait-il pas une solution d'avenir, et qui le restera longtemps ? toutes les potentialités de ce vecteur énergétique, qui renferme trois fois plus d'énergie que l'essence, mais simplement de rappeler à quelles conditions et pour quels usages l'hydrogène pourrait être une réponse adaptée aux grands enjeux énergétiques et climatiques. Tout d'abord, l'hydrogène ne sera une solution durable que si sa production est décarbonée. Nous en sommes encore très loin, puisque, aujourd'hui, 94 % de l'hydrogène produit en France l'est France l'est à partir d'énergies fossiles et que cette production représente environ 3 % des émissions nationales de CO2. Et, quand l'hydrogène est produit par électrolyse de l'eau, encore faut-il s'assurer que l'électricité est elle-même produite à partir de sources bas carbone, qu'il s'agisse du nucléaire ou d'énergies renouvelables. En découle une autre question : celle de la compétitivité économique de cet hydrogène décarboné par rapport à l'hydrogène obtenu à partir d'énergies fossiles. Même si les technologies d'électrolyse progressent rapidement, les coûts varient encore du simple au double lorsqu'il s'agit de produire de grandes quantités, l'hydrogène propre n'étant aujourd'hui compétitif que pour certains usages industriels de niche. Madame la secrétaire d'État, le Gouvernement s'est fixé comme objectif d'incorporer 20 % à 40 % d'hydrogène décarboné dans l'hydrogène industriel d'ici à 2028, en mobilisant notamment 100 millions d'euros pour des appels à projets, et en instaurant une traçabilité de l'hydrogène décarboné. Mais ces mesures sont-elles vraiment à la hauteur du changement d'échelle espéré ? En matière de stockage, le potentiel de l'hydrogène, notamment pour assurer le stockage saisonnier de l'électricité et répondre à l'intermittence des productions renouvelables, ce domaine également, il faut rappeler que l'hydrogène est en concurrence avec d'autres technologies- je pense aux stations de transfert d'énergie par pompage, ou encore aux batteries, dont les coûts ne cessent de baisser. À moyen terme terme au moins, le stockage par hydrogène ne pourra répondre qu'à des situations très spécifiques, notamment dans les zones non interconnectées, avec des réseaux isolés ou présentant un fort taux d'intégration d'énergies renouvelables intermittentes. De même, en matière de mobilité, l'hydrogène peut constituer l'une des solutions pour réduire nos émissions. Mais il viendra en complément des autres solutions que sont l'hybridation, la mobilité électrique et le bioGNV, et seulement pour les usages où il est le plus adapté, en particulier pour les transports lourds ou pour les flottes de véhicules, par exemple pour la livraison en milieu urbain. Sur le segment des voitures particulières, l'électrification et le biogaz présentent, me semble-t-il, plus d'avantages que l'hydrogène, dont les surcoûts à l'achat et à l'usage- il faut toujours penser aux prix supportables pour les ménages et les familles ! -, dès lors que l'on voudrait s'approvisionner en hydrogène décarboné,

La manière dont vous entendez favoriser concrètement le développement d'une gamme de véhicules lourds et accompagner les collectivités dans la mise en place de flottes territoriales n'apparaît pas clairement : mais sans doute pourrez-vous nous en dire davantage à ce propos dans quelques minutes, de l'hydrogène ou des autres vecteurs énergétiques, il nous faut raisonner sans, sans idéologie : la transition énergétique passera passera par une multitude de solutions, dont il importe de bien mesurer les avantages, les inconvénients, et surtout les coûts complets. La parole

Vous l'avez tous dit, le Gouvernement, sous l'égide de Nicolas Hulot, a publié, le 1 juin 2018, une feuille de route pour l'hydrogène. Il a présenté un plan ambitieux pour que l'hydrogène puisse prendre toute sa place dans la transition énergétique. Le fil directeur, c'est l'idée d'accompagner l'innovation,

Ce plan repose sur trois axes : décarboner les usages existants de l'industrie, développer des usages pour la mobilité propre, et, à moyen terme, utiliser l'hydrogène dans le système énergétique. L'année 2019 sera bien celle de l'amorçage, qui permettra d'avancer- je peux vous rassurer sur ce point.

Les volumes d'hydrogène actuellement consommés sont importants, et la réduction de ces émissions est un enjeu majeur. Notre objectif est d'amorcer le déploiement de la technologie de l'électrolyse en France, pour changer d'échelle en faisant baisser les coûts et en soutenant la montée en performance des électrolyseurs.

Cela concerne notamment les petits industriels, dans les secteurs de la chimie, de la verrerie, dont les besoins sont relativement limités et auxquels l'hydrogène est aujourd'hui livré par camion. Ce n'est pas pour autant un marché facile à développer, parce qu'il faut convaincre l'industriel d'investir dans un électrolyseur pour plusieurs années, ce qui suppose un changement de pratiques. Pour atteindre les objectifs de décarbonation de l'État, un appel à projets sera bientôt lancé pour le déploiement et l'industrialisation de la production décarbonée d'hydrogène, en complémentarité avec les outils existants relatifs à la démonstration et à la recherche. Une aide de l'État permettra donc de surmonter la barrière que représente l'investissement prévu dans le

le comité stratégique de filière sur les énergies renouvelables s'est emparé de la question de l'hydrogène et formulera prochainement des propositions en ce sens.

L'hydrogène est en effet l'une des solutions clés pour développer les mobilités propres, en complémentarité avec le biogaz et les batteries ; plusieurs d'entre vous en ont parlé. L'hydrogène présente trois avantages majeurs pour les usages intensifs et dans les transports lourds. Le temps de recharge est réduit- trois minutes -, très comparable à un plein d'essence,

axe du plan Hydrogène concerne les perspectives de stockage des énergies renouvelables. Vous l'avez dit, l'hydrogène produit par électrolyse est, à long terme, une solution structurante pour l'intégration des énergies renouvelables au système électrique, notamment en tant que moyen de stockage massif des énergies intermittentes et de stockage massif intersaisonnier. L'électricité est ainsi stockée sous forme d'hydrogène qui peut être soit valorisé directement, soit injecté dans les réseaux gaz, soit injecté sous forme de méthane de synthèse dans les réseaux gaz après recombinaison avec du CO2 par le procédé de méthanation. La complémentarité de ce procédé avec la méthanisation classique a été évoquée. Les réseaux de gaz représentent donc un moyen de stockage de l'électricité et l'hydrogène Les réseaux de gaz représentent donc un moyen de stockage de l'électricité et l'hydrogène permettant d'optimiser et de mutualiser le système énergétique. Par ailleurs, les besoins de flexibilité émergent d'ores et déjà dans les zones ayant des taux de déploiement d'énergies renouvelables intermittentes importants. Je pense en particulier aux

Ces interactions entre électricité et gaz offrent de nouvelles perspectives, à moyen et à long termes, pour ces deux secteurs, mais aussi pour l'industrie. Le « » constitue une opportunité de décarboner les réseaux de gaz et encourage le développement des énergies renouvelables électriques-

Nous allons lancer des expérimentations dans ces zones non interconnectées pour y développer au plus vite l'hydrogène et les électrolyseurs. De plus, plus, afin de préparer l'arrivée du procédé « », nous avons confié aux gestionnaires d'infrastructures gazières- GRTGaz, GRDF et Storengy -la mission de déterminer les conditions techniques et économiques, dont celles qui sont relatives à la sécurité, évidemment fondamentales. Le rapport intermédiaire confirme d'ores et déjà les premières conditions d'injection envisageables, avec un rapport final prévu cet été. Au-delà des axes sectoriels que je viens de vous présenter, nous travaillons avec les différents acteurs de la filière à des engagements pour la croissance verte qui devront permettre, d'abord, de valoriser et de faire connaître les actions en cours de la filière française de l'hydrogène, dite « Équipe de France Hydrogène », car il est très important de valoriser l'action menée en France et à l'international, ensuite, de faciliter le déploiement de la filière hydrogène avec un travail sur les freins à lever- c'est ce qui a lieu dans le comité stratégique de filière -, enfin, d'avoir des engagements concrets des acteurs français de l'hydrogène, en complément à ceux de l'État pris dans le plan Ce travail encourage les acteurs de l'hydrogène à se regrouper pour faire émerger les nouveaux usages, les technologies, les produits et les services indispensables à la réussite du plan.

En conclusion, le plan Hydrogène n'est qu'un début. Il traduit une ambition. Il n'est pas figé, il n'est pas non plus fini, car nous devrons le faire vivre collectivement, avec tous les acteurs. C'est un accélérateur de la transition écologique, dans l'industrie, dans l'énergie

La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande du débat dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'aimerais pouvoir vous dire qu'il s'agit du dernier débat sénatorial sur la fracture numérique auquel nous participons aujourd'hui. Malheureusement, nous savons tous que ce n'est pas le cas. Le Sénat continuera d'aborder cette question, d'abord parce qu'il a chevillé au corps tout ce qui a trait à l'aménagement du territoire, mais surtout, parce que, malgré les efforts réels des gouvernements qui se succèdent, nous sommes face à une révolution qui, comme le chemin de fer en son temps, se déroulera sur plusieurs décennies. Comme le chemin de fer, donc, comme tout progrès en somme, le numérique entraîne son lot d'externalités, tantôt positives, tantôt négatives. Et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui à mesure qu'une technologie se développe, des usages se développent eux aussi. Puis ce sont les comportements qui évoluent : e-commerce, télétravail,, télémédecine, tous ces phénomènes ont une incidence directe sur l'aménagement du territoire.

Voilà la genèse de ce débat sur la fracture numérique et les inégalités d'accès aux services publics. Pour le groupe Les Républicains, qui en est à l'origine, il paraît plus que nécessaire, à l'aune de ce rapport, que le Gouvernement dévoile sa stratégie.

Le rapport commence par cette affirmation : au moment où les transformations de l'organisation de l'État, mais également des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, ou encore du système de santé, se traduisent par un recul de sa présence au plus près des usagers, cette révolution numérique offre de nouveaux moyens d'accès aux services publics. Certains répondront avec malice que le numérique n'est pas uniquement l'une des conséquences de la restructuration de l'État, mais qu'il peut être aussi l'une de ses causes. Ne sachant pas qui, de l'oeuf ou de la poule, est arrivé en premier, je ne trancherai pas. Quoi qu'il en soit, l'apport de la dématérialisation à l'amélioration de l'accès aux services publics est incontestable. Pour s'en convaincre, je donnerai En 2017, plus de 20 millions de foyers fiscaux ont déclaré leurs revenus en ligne, soit 2,4 millions de foyers fiscaux supplémentaires par rapport à 2016. 90 % des utilisateurs se déclarent satisfaits de ce service. Enfin, les services numériques des administrations sont jugés en avance ou au même niveau que les services des entreprises privées par 70 % des Français. Je prendrai maintenant un cas pratique. Aux termes d'une étude du ministère des solidarités et de la santé, la dématérialisation s'est révélée un facteur d'amélioration de l'accès à la prime d'activité, avec un taux de recours élevé, estimé à 73 %, dépassant de 23 % les projections initiales. Le rapport détaille enfin sous quelles conditions la dématérialisation est une avancée pour l'accès aux services publics : elle doit s'inscrire dans une démarche large portant sur les simplifications possibles des procédures administratives et sur les capacités qu'offre la technologie pour repérer et résoudre les situations de non-recours. J'en arrive au deuxième grand point du rapport précité. Il existe des fractures sociales et territoriales qui aggravent, la dématérialisation, les inégalités d'accès aux services publics. Qui peut croire que la dématérialisation est indolore lorsqu'on est situé en zone blanche ? Je ne reprendrai pas à mon compte la liste des communes concernées, identifiées par arrêté, car je crois le problème beaucoup plus profond. Les zones blanches et ces quelques communes officielles ne sont que la face émergée de l'iceberg. Une statistique me semble éloquente pour rendre compte de la fracture territoriale. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, plus d'un tiers des habitants n'ont pas accès à un internet de qualité, ce qui représente près de 75 % des communes de France et 15 % de la population. Bien sûr, les territoires ruraux et les territoires ultramarins arrivent en tête. Le rapport du Défenseur des droits ne s'arrête pas à cela. Bien qu'elle n'ait pas de lien direct avec la fracture territoriale- quoique -, il rappelle que la dématérialisation accroît les inégalités du fait de l'inaccessibilité financière aux abonnements à internet et au matériel informatique : ordinateurs, imprimantes, scanners ou smartphone. La dimension sociale rejoint souvent la dimension territoriale. Ceux de nos concitoyens qui éprouvent le plus de difficultés résident souvent dans les territoires enclavés ou insulaires. Enfin, les inégalités d'accès aux services publics se nourrissent des obstacles techniques, voire du défaut de conception ou d'ergonomie des sites et des procédures dématérialisées, sans oublier les problèmes liés au paiement dématérialisé. Si les sources de ces inégalités sont nombreuses, les publics victimes de ces difficultés sont, eux aussi, très nombreux et variés. On parle alors de fracture sociale et culturelle. Autre statistique éloquente du document susvisé, le taux de connexion à internet varie de 54 % pour les non-diplômés à 94 % pour les diplômés de l'enseignement supérieur.

Quel lien y a-t-il entre dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics ? La réponse a été rapide à trouver et je la résumerai en une phrase oui, la dématérialisation des démarches administratives crée des inégalités d'accès aux services publics, mais ces inégalités sont le fait de la fracture numérique et non de la technologie en elle-même. Oui, il est Oui, il est possible de développer du numérique inclusif ; le seul tort de la technologie est de donner une opportunité à l'administration de masquer son approche budgétaire et comptable en invoquant la modernité et la qualité du service public ; mais rien de plus Les administrations ont, elles aussi, une petite part de responsabilité, mais, à leur décharge, elles évoluent dans un cadre budgétaire contraint, et le développement des téléprocédures a été un véritable mirage comptable pour elles. Pensons que, depuis 2013, a eu lieu le choc de simplification, puis le programme de transformation de l'administration, baptisé « Action publique 2022 »,

C'est indiscutable, l'administration a pris la mesure des inégalités entraînées par la dématérialisation. Elle apporte des réponses à la fracture sociale qui accroît les inégalités. Je pense aux inégalités liées à l'accessibilité financière au numérique, ou encore aux usages, notamment pour les personnes âgées. Mais je ne crois pas que la fracture territoriale, elle aussi source d'inégalités dans l'accès aux services publics, soit pleinement appréhendée. Chaque mois, de nouvelles téléprocédures apparaissent, de telle sorte que la fracture territoriale devient de plus en plus insupportable. Alors oui, il est loisible, pour le Gouvernement, de prendre les mesures d'urgence, notamment sur recommandation du Défenseur des droits. Mais si la fracture sociale et culturelle peut trouver des réponses par le biais d'un accompagnement- favoriser l'usage d'un identifiant unique, renforcer la formation initiale et continue des travailleurs sociaux et des agents des agents d'accueil des services publics à l'usage numérique, créer une clause de protection des usagers en cas de problème technique -, la lutte contre la fracture numérique ne peut faire l'économie de mesures beaucoup plus profondes. Je suis sensible, par exemple, à la proposition du Défenseur des droits de voir adopter des dispositions législatives.

le secrétaire d'État, que peut-on faire pour la téléphonie mobile depuis le lancement du ? Voilà quelques jours, le Président de la République, sous la pression des élus exaspérés, annonçait vouloir mettre la pression à son tour sur les opérateurs. Cette déclaration correspond-elle à un changement de braquet ? Doit-on s'attendre à des changements sur le statut de zone fibrée ? Qu'attend le Gouvernement pour rouvrir le guichet du plan France très haut débit ? Enfin, ultime question, pendant encore combien de temps allons-nous accepter que des principes aussi élémentaires que celui de l'égalité devant le service public soient bafoués ? La parole

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

Nombreux sont ceux qui ont l'impression de ne pas parler le même langage que l'administration et qui se découragent devant la multiplicité et la complexité des démarches, allant parfois jusqu'à renoncer aux droits qui leur sont dus. Nombreux sont ceux qui bénéficieront de cette formidable possibilité de réaliser leurs démarches administratives à toute heure du jour ou de la nuit, sans attendre une RTT ou poser une demi-journée Mais c'est une lame à double tranchant. La technologie numérique ne doit pas être un outil d'amoindrissement du service public et d'économies de bouts de chandelle au détriment des plus fragiles. L'enquête du Défenseur des droits sur les impacts de la numérisation des services publics que celle-ci ne rend pas service à ceux qui en auraient le plus besoin lorsqu'elle se substitue à l'accueil humain. Elle revient alors à ériger un nouveau fossé entre l'administration et les citoyens. Numérisation ne doit pas rimer avec désertification, car internet n'est qu'un outil qui ne peut se substituer intégralement à l'humain. Tel est le cas, tout d'abord, parce que 8 % des Français, soit plus de 5 millions de nos compatriotes, n'ont pas accès à internet, mais aussi parce que des millions d'autres ne sont pas suffisamment familiarisés avec cet outil ou ne sont pas en mesure de l'utiliser seuls. Aussi, la numérisation progressive de l'administration doit être accompagnée par des agents répartis le plus finement possible sur le territoire. Quoi de plus efficace, pour ce faire, que les mairies de nos 36 000 communes, qui sont le maillage le plus fin possible du territoire ?

ou pour ceux qui ont besoin d'être orientés. C'est aussi le travail qu'ont mené les équipes de la mission Société numérique, toute l'année dernière, en collaboration avec les départements et les régions de France : déterminer, en toute finesse, qui sont ces oubliés du numérique. Quels sont ceux qui n'ont pas le réseau ? Quels sont ceux qui n'apprendront jamais ?

soit parce qu'ils n'en maîtrisent pas les usages. En parallèle, la dématérialisation des services publics, si elle répond à un besoin d'efficacité et d'efficience que nul ne conteste, ne doit pas entraîner une déresponsabilisation des pouvoirs publics renvoyant à la sphère associative l'accompagnement des usagers. Le rapport récent sur le sujet du Défenseur des droits sonne l'alerte et relève très justement le risque de privation de droits liée à la déconnexion ou à l'illectronisme des usagers. Il faut donc conserver une présence physique du service public, car elle est conforme au principe constitutionnel d'égalité devant le service public. L'association Emmaüs Connect, très impliquée dans l'inclusion des plus fragiles, estime qu'il faudrait un milliard d'euros, sur sept ans, pour financer l'inclusion numérique, tandis que le Gouvernement prévoit de mobiliser à peine 100 millions d'euros.

les, ou villes sûres et intelligentes, comme Angers, va transformer profondément nos services publics par la numérisation généralisée. Il faudra bien sûr veiller à l'inclusion sociale et technologique des habitants. Aussi la numérisation pose-t-elle également la question de la souveraineté, ce qui avait bien été mis en exergue par le rapport parlementaire de M. Luc Belot, paru en avril 2017. En effet, la mise à disposition de- données stratégiques utilisées par des applications en tous genres -pourrait, à terme, déposséder les collectivités de leurs services publics locaux. Devant cette nouvelle menace de fracture numérique,

de l'inclusion numérique des plus éloignés est une priorité du Gouvernement. Une méthode que nous avons adoptée très tôt part du principe qu'aucune solution venant d'en haut ne peut fonctionner. Pendant près d'un an et demi, nous avons travaillé avec l'Assemblée des départements de France et avec de nombreux présidents de département, qui sont venus eux-mêmes

Quand on ne sait pas utiliser internet, on est moins informé. Quand on ne sait pas utiliser internet, on communique moins avec son entourage. Quand on ne sait pas utiliser internet, c'est la double peine, et on paye tout plus cher : statistiquement, dès que les Français achètent un objet d'une valeur supérieure à 100 euros, ils comparent toujours en ligne.

par un meilleur accès aux soins, notamment grâce à la télémédecine, dans toutes ses composantes, de la téléconsultation à la téléexpertise. Les ambitions de la France en la matière sont immenses, de même que ses atouts, avec un système de santé de qualité reconnu dans le monde entier. Mais le déploiement de la télémédecine se heurte encore à plusieurs difficultés, notamment, au manque d'efficience du réseau certains territoires. Dans le Grand Est, par exemple, nous avons lancé un plan massif visant à doter de la fibre optique, d'ici à 2023, chaque habitation de la région. Au-delà du déploiement du très haut débit, les professionnels de santé éprouvent néanmoins des difficultés à s'organiser. 35 % d'entre eux disent connaître correctement les technologies de santé connectée. Ils ont besoin de plus d'ingénierie, de plus d'accompagnement et de plus de formation pour mettre en place les outils et les organisations nécessaires et ainsi faire profiter pleinement leurs patients des atouts du numérique.

de l'avenant : « Tout assuré, quel que soit son lieu de résidence, et tout médecin, quelle que soit sa spécialité, pourra y recourir. » Je considère toujours cette mesure comme une réponse, parmi d'autres, au phénomène de désertification médicale. Toutefois, des freins semblent exister. La CNAM a récemment annulé le remboursement des consultations effectuées par des patients patients n'étant pas domiciliés à proximité du médecin qui assure la téléconsultation. Quel est l'état d'esprit du Gouvernement sur ce sujet, et quelles pistes sont envisagées pour lever ces freins ?

la téléconsultation, qui rend accessible un médecin à une personne à un moment où, physiquement, celui-ci n'aurait pas pu être près d'elle. Cela évite au patient de devoir parcourir une distance qu'il n'aurait peut-être pas pu franchir seul et met à sa disposition, près de chez lui,

que le médecin consulté était trop éloigné. En effet, pour cet an 1 de la téléconsultation, nous avons souhaité qu'elle soit réservée à la relation entre un médecin généraliste et un patient qu'il a l'habitude de recevoir ou qu'il pourrait avoir l'habitude de recevoir.

nous dénaturerions le fameux lien humain dont nous parlions précédemment. Une téléconsultation avec des humains, une téléconsultation remboursée, une téléconsultation reconnue par l'Ordre des médecins comme étant une consultation médicale de qualité, voilà l'ambition ! Rappelons que 2019 est l'année du remboursement de toutes ces téléconsultations.

Merci, monsieur le ministre,

Dans les territoires à faible densité de population, on ne peut plus se contenter de courir sans cesse derrière la technologie, avec cinq ou dix ans de retard ! Êtes-vous prêt, monsieur le ministre, à inverser la logique qui a creusé ces inégalités territoriales quand on aurait dû les réduire ? Êtes-vous prêt, à l'avenir, à avancer au même rythme

J'étais moi-même dans le Cantal, il y a quelque temps, auprès d'un ami cher, pour évoquer le déploiement du numérique, mais aussi de la téléphonie mobile.

sans aucun doute, l'un des défis majeurs de notre époque ; une chance, autant qu'un risque. Il représente une chance pour chacun d'accéder à de nouveaux services, à de nouvelles technologies, de gagner du temps, de rester en contact avec l'autre, une opportunité pour les services publics, qui doivent se moderniser. Certains pays, comme l'Estonie, y parviennent très bien. C'est un enjeu politique et social pour simplifier la vie des citoyens et améliorer leur quotidien, comme pour permettre à l'État de faire des économies.

Le Sénat n'a pas manqué d'alerter les gouvernements successifs sur les risques de fracture territoriale et sociale dans notre pays. La réorganisation des services publics et les réformes territoriales additionnées à l'absence de politique d'aménagement du territoire ont été vécues douloureusement, notamment

Les services de l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS, sont injoignables et une simple erreur matérielle dans la demande nécessite un renouvellement total et non une rectification simple à la charge de l'administration. C'est inadmissible Pour conclure, nous ne pouvons rester sur un constat d'échec. Fort heureusement, ça bouge dans nos départements ! En Charente-Maritime, nous avons pour ambition de couvrir 100 % du territoire en fibre optique d'ici à 2022, la désertification médicale fait l'objet d'un accompagnement des zones les plus isolées et les maisons de services au public sont au sont au plus près des citoyens. Nous avons une obligation de réussite. Monsieur le secrétaire d'État, la verticalité a ses limites et peut empêcher de voir l'horizon. Au Sénat, nous sommes la voix des territoires, merci de nous entendre

de confirmer qu'une grande partie des personnes qui ne maîtrisent pas le numérique aujourd'hui pouvaient être formées en dix à vingt heures aux usages de base : se connecter à internet ou utiliser un et un mot de passe. C'est pour cela que votre département a mis en place, avec Pôle emploi,

considérable dans notre quotidien. Les infrastructures, leur implantation et leur accessibilité sont une problématique que nous abordons souvent dans cet hémicycle, afin de réduire ce que l'on appelle la fracture numérique. Se posent également aujourd'hui, de façon systématique, la question des usages ainsi que celle de l'inclusion numérique. Jeudi dernier, vous étiez en déplacement à Labège, près de Toulouse, pour échanger avec des acteurs impliqués dans ce domaine dans le cadre d'une étape du Tour de France des oubliés du numérique, visant à identifier les problématiques, mais aussi les initiatives remarquables en la matière.

Dans mon département, la Gironde, des assises des solidarités numériques étaient organisées au mois de décembre dernier. Dédiées au développement social, elles avaient pour objectif d'apporter aux collectivités et aux associations les outils nécessaires pour tendre vers un usage du numérique facilitant le lien social. Alors que l'administration française migre de plus en plus vers des services numériques, alors qu'une directive européenne introduit l'obligation, pour les sites appartenant à une instance publique, d'être accessibles aux personnes handicapées,

Je voudrais plutôt revenir sur un autre aspect de cette fracture : les difficultés liées à l'usage, que certains dénomment l'illettrisme numérique, ou l'illectronisme. Aujourd'hui, 20 % de nos concitoyens ne savent pas utiliser internet, soit 13 millions de personnes, dont plus de la moitié ne se connecte jamais. Le coût de l'équipement est aussi un frein : selon une étude d'Emmaüs, 35 % des personnes vivant sous le seuil de pauvreté n'utilisent jamais internet. Alors que le mot d'ordre est la dématérialisation des services publics, cela pose une sérieuse question d'accès aux droits dans un nombre croissant de secteurs- la sécurité sociale, la recherche d'emploi, les déclarations PAC, pour les agriculteurs, l'orientation universitaire avec Parcoursup -, voire un problème d'accès à la démocratie, puisque même l'organisation du grand débat se fait essentiellement internet. La réforme de la justice, notamment, est une source d'inquiétude de ce point de vue, puisqu'elle comporte un large volet consacré à la dématérialisation de l'accès à la justice. En remettant en cause l'accès direct au juge, on fait reposer la garantie du respect des droits fondamentaux des citoyens sur le postulat d'un accès universel à l'outil informatique.

Aujourd'hui, force est de constater que les réponses ne sont pas à la hauteur des besoins. Ainsi, le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté prévoyait, certes, des bornes d'accès au droit dans des lieux d'accueil de personnes en grande difficulté, mais pas l'accompagnement nécessaire pour que l'accès à ces bornes soit effectif. De même, le Gouvernement présentera prochainement une liste d'une dizaine de lieux de médiation numérique pour conseiller et former les populations les plus éloignées d'internet, soit même pas un par grande région Pour que les progrès techniques soient véritablement synonymes de progrès social et non source d'une exclusion supplémentaire, le volontarisme des pouvoirs publics doit être identique à celui qui avait été déployé pour combattre l'illettrisme.

J'y suis particulièrement sensible et attentif : je représente un territoire, la Vienne, dont les habitants sont directement concernés par les fractures territoriales, la fracture numérique et la fermeture ou l'éloignement des services publics. Lorsque l'on Lorsque l'on évoque la fracture numérique, s'agissant de l'accès aux services publics, on pense spontanément à la dématérialisation des démarches et des formalités administratives. De très nombreux services sont concernés, tant pour les particuliers que pour les professionnels et les associations.

la qualité trop souvent aléatoire des réseaux numériques dans certains territoires, et- ce n'est pas moins problématique -la part non négligeable de la population qui reste réfractaire à cet outil. Les troubles subis dans notre pays doivent faire comprendre à tous que les plus mal lotis, dans la France périphérique, doivent aussi être écoutés. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, jusqu'où le Gouvernement projette-t-il d'aller en matière de dématérialisation, tout particulièrement en ce qui concerne les fonctions régaliennes de l'État que sont la police et la justice ? Le passage au tout-numérique reste éloigné et une approche humaine suppose des solutions complémentaires. Le Défenseur des droits recommande de préserver plusieurs modalités d'accès aux services publics, afin qu'aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée. Cela me semble indispensable. Quelles synergies envisagez-vous entre numérique et points de rencontre physiques, en particulier avec le réseau des MSAP ? Ces synergies doivent permettre de garantir l'accès aux services publics aux Français porteurs de différents handicaps. Comment intégrez-vous cette réalité ? La parole

de téléphonie ou d'accès à internet. Or une partie des territoires est encore, nous l'avons déjà dit, mal équipée, voire sous-équipée, rendant ces conditions difficiles, voire impossibles. Dans certaines communes rurales d'Occitanie, notamment dans les Hautes-Pyrénées, le manque de couverture réseau pour les téléphones portables et les débits trop faibles d'accès à internet constituent une réelle fracture numérique pour un grand nombre de nos concitoyens. L'aménagement des réseaux en très haut débit des Hautes-Pyrénées doit être finalisé d'ici à cinq ans. Cependant, on peut douter que les équipements soient totalement opérationnels en un laps de temps si court. C'est une fracture à la fois sociale et territoriale. En effet, les projets de fermeture ou d'éloignement des services publics traditionnels, comme les trésoreries ou les bureaux de poste, ainsi que la disparition de certaines compétences municipales, comme l'instruction des cartes nationales d'identité et des passeports, ajoutent de nouvelles difficultés. C'est aussi une fracture sociale qui frappe surtout nos concitoyens les plus fragiles, les personnes âgées ou au chômage, qui ne sont pas toujours à l'aise avec les nouveaux usages numériques ou qui n'ont pas toujours les moyens de posséder un ordinateur et de se former à son utilisation. Le désert numérique, qui s'ajoute très souvent à un désert médical, aggrave une inégalité territoriale totalement inconcevable et un sentiment d'abandon chez nombre de nos concitoyens. Monsieur le ministre, le tout-numérique ne peut être l'unique solution. Si la préservation de l'accès aux services publics, y compris dans les zones rurales les plus reculées, constitue bien une priorité pour le Gouvernement, il lui faudra conserver une diversité d'approches. Que comptez-vous faire alors pour le maintien, le développement et l'évolution des autres moyens d'accès aux services publics que le numérique ?

l'importance de ma question, la diversité des approches des services publics autres que le numérique. Vous avez parlé de l'humain. Mais je tiens quand même à rappeler- je rejoins là ma collègue Anne-Catherine Loisier -que, dans mon département,

le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, si la France est une République indivisible, on ne peut pas dire que l'accès au numérique soit homogène dans notre pays, vous l'avez rappelé. Il entraîne une véritable inégalité en matière d'accès aux services publics. Pourtant, que l'on soit dans le Perche, les Cévennes ou le Mantois, on a besoin à la fois de l'un et de l'autre. Depuis quelques années, nous empruntons le chemin de la fin de l'hyperproximité des services publics. Nous avons dû nous adapter aux fermetures sèches, aux mutualisations et rationalisations de certains de nos services. Nous en connaissons les raisons ; je ne les évoquerai pas. Pour réduire la fracture territoriale, nous avons fait le choix de dématérialiser certaines fonctions. Cette orientation stratégique n'est pas dénuée de fondement, car elle permet de compenser, en partie tout du moins, le départ de certains services publics. Le gain potentiel pour l'usager comme pour les services publics peut sembler immense. Je souhaite tout de même insister sur le caractère « potentiel », car, en l'état actuel des choses, l'accès au numérique est insuffisant. Ne perdons pas de vue plusieurs notions essentielles : le principe de continuité du service public, le principe de l'égalité devant le service public et, enfin, les principes d'adaptabilité et de mutabilité. Former, accompagner et simplifier doivent être autant de pistes auxquelles il convient de réfléchir en tenant compte des spécificités de nos territoires et de leurs habitants. Enfin, ayons en tête, monsieur le secrétaire d'État, que le numérique ne doit pas être un palliatif à la disparition des services publics dans nos territoires.

toujours trop présente, sans que cela se fasse évidemment au détriment du service de proximité ? Deuxièmement, on connaît l'importance de la qualité d'adressage d'une commune, qui est fondamentale pour l'aménagement du territoire. Or la fracture numérique est parfois due à un manquement

nous ne devons jamais réorganiser territorialement sans nous poser la question de l'accessibilité réelle et physique à un être humain. Quand il s'agit de fermer une trésorerie- et nous en fermerons

je ne pense pas que la relation entre l'administré et l'administration puisse se faire au travers d'un écran. D'ailleurs, de ce point de vue, la sémantique est importante.

Cependant, malgré la poursuite du déploiement et l'abondement des crédits, le dispositif est gelé jusqu'à la mi-2019 à la demande des opérateurs, qui s'interrogent sur l'efficacité de certaines MSAP. Toutefois, il existe des enjeux immédiats et des dispositifs à mettre en place à court terme tant il est évident que l'accès aux services publics, sous une forme ou une autre, est un enjeu de notre société et une préoccupation de nos concitoyens.

Comment et quand les collectivités locales engagées dans la gestion des MSAP vont-elles être aidées financièrement ? Enfin, le financement par l'État du déploiement de la fibre est gelé, alors qu'il reste un nombre de foyers important à desservir. Est-ce temporaire ou définitif ? Dans un autre domaine, le dispositif mis en place par l'État pour résorber les zones blanches de téléphonie mobile reste très limité par le nombre de sites possibles au regard de l'ampleur de la problématique- cette question a également été évoquée précédemment. En outre, il est contestable sur la méthode : les collectivités sont parfois obligées de financer des études alors que les opérateurs disposent d'informations précises, mais ne veulent pas les communiquer pour des raisons de concurrence. Quelles mesures envisagez-vous de prendre, afin d'accélérer

L'Assemblée des départements de France est notre premier partenaire sur le sujet. Aujourd'hui, tous les départements ont compris que l'inclusion numérique était le nouveau pilier du chapitre concernant l'action sociale territoriale et qu'il était absolument nécessaire

Le 14 janvier 2018, un accord a été signé entre l'État, l'Arcep et les quatre opérateurs de téléphonie mobile. Par ce biais, l'aménagement numérique du territoire devient prioritaire dans les conditions d'attribution des fréquences. Cet accord est contraignant pour les opérateurs, qui vont devoir, d'une part, équiper l'ensemble des sites de téléphonie existants en 4G et, d'autre part, construire d'ici à trois ans 5 000 sites mobiles chacun, sites parfois mutualisés, afin d'accélérer la cadence de déploiement des réseaux mobiles. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire part des résultats de cet accord à date ? Comment votre ministère envisage-t-il le déploiement de la 5G dans ces territoires, alors que les fréquences seront attribuées dans les prochains mois ? Les territoires de montagne devront-ils encore attendre une décennie pour y avoir accès ?

ce débat a naturellement une résonance particulière dans le contexte actuel. L'exaspération exprimée au cours des dernières semaines, face aux inégalités vécues et perçues dans les territoires, se nourrit aussi de la fracture numérique. L'absence d'accès au numérique est aujourd'hui ressentie, par nos concitoyens, comme une forme de déclassement et une véritable injustice, à juste titre. Ce sentiment devient de plus en plus violent avec la généralisation des services en ligne, dans tous les domaines. C'est la double peine Je reviens à la question spécifique de la dématérialisation des services publics et de l'ambition portée par l'exécutif. Comme l'a rappelé le Défenseur des droits, « la mise en oeuvre des politiques publiques de dématérialisation se doit [ ...] de respecter les principes fondateurs du service public l'adaptabilité, la continuité et l'égalité devant le service public », ce qui nécessite une connexion internet de qualité et l'accès à des équipements informatiques. Or ces deux conditions évidentes ne sont pas réunies partout- les chiffres en la matière ont été rappelés au cours du débat. Face à ce constat, quelles réponses apporter ? L'amélioration significative de la couverture numérique du territoire et de l'accès des Français au très haut débit, tant fixe que mobile, reste la condition pour lutter contre la fracture numérique. Faut-il rappeler qu'en moins de dix ans seulement, le déploiement des technologies de l'information et de la communication est devenu une composante essentielle du développement et de la compétitivité des territoires ? Alors oui, monsieur le ministre, monsieur le

Dans le contexte actuel, la non-réalisation ou un nouveau report des objectifs fixés pourrait avoir des conséquences encore bien pires que celles de l'augmentation inconsidérée de la taxe carbone. En janvier dernier, devant les maires, le Président de la République a indiqué vouloir mettre la pression sur les opérateurs pour que le déploiement se fasse au bon rythme. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que les engagements seront bien tenus, à l'horizon de 2020 pour le haut débit et de 2022 pour le très haut débit,

Quels nouveaux leviers l'exécutif entend-il actionner pour contraindre les opérateurs ? Pour les zones qui ne pourront pas techniquement avoir accès à la fibre jusqu'au domicile en 2020, le Gouvernement a ouvert, à compter du 1 janvier 2019, un guichet « cohésion numérique des territoires Cette enveloppe est-elle réellement à la hauteur des besoins ? C'est une véritable question ! Outre la couverture numérique des territoires, la dématérialisation des services publics devra nécessairement s'accompagner d'une attention particulière portée à la capacité des familles à s'équiper en matériel informatique. En 2017, 19 % de la population ne possédait pas d'ordinateur, le prix du matériel étant le premier frein. Le sujet de l'obsolescence programmée des appareils et de ses conséquences, tant économiques qu'écologiques, doit également être soulevé par l'État, de même que l'accessibilité et les conditions de résiliation Autre danger, la dématérialisation de l'intégralité des services publics en 2022, très largement évoquée dans cet hémicycle aujourd'hui, ne peut se résumer à compenser la disparition des services publics sur certains territoires

mes chers collègues, nos concitoyens demandent avant tout une présence physique des services publics dans les territoires. Prenons pour exemple la télémédecine : si celle-ci représente un vecteur important d'amélioration de l'accès aux soins, en particulier dans les zones sous-équipées, elle ne saurait se soustraire aux actes médicaux classiques et à la présence, sur nos territoires, la dématérialisation des services publics pourra fonctionner seulement si elle s'accompagne d'un effort de simplification et de rationalisation. À ce titre, la proposition du Défenseur des droits d'instaurer un identifiant unique me paraît intéressante et prioritaire. Simplifions la vie de nos concitoyens ! Enfin, si l'État s'est engagé à fournir un nouvel effort financier en faveur des réseaux d'initiative publique portés par les collectivités en décembre dernier, ce dont je me félicite,